considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, de

Ce budget, lors de sa planification, traduisait le choix d'un système de santé renforcé et empreint de justice pour mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et de nos professionnels de santé. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale- vous le rappeliez lundi dernier, monsieur le ministre -était un texte d'engagement et d'investissement pour notre système de santé, une première pierre à l'effort de refondation. Très concrètement, pour les Français qui nous écoutent, ce projet de loi, dans sa version originelle, permettait de trouver plus facilement un médecin traitant, d'attendre moins longtemps aux urgences, de trouver une aide à domicile pour son parent âgé ou en situation de handicap, de bénéficier d'un mode d'accueil pour son enfant, d'être mieux soutenu en tant que famille monoparentale et, enfin, d'effectuer plus facilement ses déclarations Urssaf en tant qu'entrepreneur. J'aimerais revenir sur deux mesures phares proposées dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. La première est le renforcement du virage préventif, qui trouve une traduction concrète dans la mise en place des rendez-vous de prévention aux âges clés- 20-25 ans, 40-45 ans et 60-65 ans -et dans l'accès facilité à la contraception d'urgence pour les femmes majeures,

mais aussi de diminuer le coût du recours à une assistante maternelle pour les parents. Pour autant, la majorité du Sénat n'a pas été convaincue par ce PLFSS. Si 18 amendements du Gouvernement ont été adoptés

mais aussi nous réjouir pour nos aînés, entre autres, de l'adoption de l'amendement du Gouvernement n° 1141, visant à majorer la compensation versée aux départements au titre des revalorisations prévues

également pu nous réjouir de l'adoption de l'amendement gouvernemental n° 943, qui vient transformer le système d'information des maisons départementales des personnes handicapées La stratégie d'harmonisation de 2015 a fortement contribué au déploiement d'une première phase de coordination des pratiques professionnelles, à l'automatisation des échanges avec les partenaires des MDPH, à la mise en oeuvre de projets structurants, ainsi qu'à la mise à disposition et à la fiabilisation d'indicateurs de pilotage. Mais ce modèle a atteint ses limites, et il est désormais temps de basculer vers un système d'information unique pour les MDPH. Enfin, notre groupe et les nombreux Français qui peinent à accéder aux soins peuvent se réjouir de deux améliorations. La première tient à l'adoption de l'amendement n° est étendue la condition de durée minimale d'exercice dans un cadre autre que des missions d'intérimaire pour les professionnels de santé mis à disposition auprès d'un établissement de santé en France dans le cadre d'un contrat conclu par une entreprise de travail temporaire établie à l'étranger.

Ce forfait permettra de couvrir les frais associés aux sujétions liées aux consultations effectuées dans les zones sous-dotées. Cela semble évident, mais notons que, pour garantir la diversité des territoires investis dans ce dispositif ainsi que leur représentativité,

ou encore la suppression de la dispense du ticket modérateur pour les consultations de prévention postérieures à 25 ans. Depuis plus de cinq ans, la majorité sénatoriale souhaite introduire par voie d'amendement une réforme paramétrique du régime des retraites. la clé du système est fondée sur le pilier de la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire sur notre régime de répartition. Le Gouvernement s'est engagé, pour réformer ce régime, à lancer une grande concertation, qui doit tenir compte d'un ensemble de paramètres sociétaux pénibilité, carrières interrompues, égalité femmes-hommes, travail des seniors. Tenter de résoudre les faiblesses de notre système en cherchant en priorité son équilibre financier est une approche limitative.

ce budget de la sécurité sociale, que nous qualifiions de « peu ambitieux » lors de la discussion générale, est resté plutôt fidèle à cette appréciation. Je rappelle que c'est la première fois qu'un PLFSS arrive au Sénat après une procédure de 49.3. Notre chambre sera donc la seule à débattre de ce texte Mais le 49.3 rend nos délibérations incertaines, puisque le Gouvernement aura à lui seul la charge d'écrire le texte définitif. Le rôle du Parlement en est réduit. Par ailleurs, le régime des irrecevabilités a encore restreint le débat, dans des proportions que nous jugeons excessives. Nous ne pourrons continuer dans cette voie à l'avenir. Enfin, la semaine a produit des débats parfois éloignés de la réalité légistique. En introduisant des articles sans lien direct avec une loi de financement de la sécurité sociale, le Gouvernement a contribué à égarer le sens du texte ; nous le déplorons. Il devient urgent de présenter un projet de loi de santé, qui tire les leçons de la pandémie et fixe l'engagement des collectivités territoriales dans ce domaine. Sur le fond, concernant la trajectoire financière, les inquiétudes que nous avions exprimées face à vos choix n'ont pas reçu de réponse claire. Vous présentez un budget social largement en déficit malgré nos propositions en matière de recettes, tout en n'investissant pas suffisamment dans notre système de soins, du moins pas à la hauteur des besoins. les exonérations fiscales, nous continuerons de faire des propositions utiles, appuyées sur des études telles que celle du Conseil d'analyse économique, pour supprimer les exonérations coûteuses et inutiles pour l'emploi.

Pis- les professionnels de santé ont du mal à le croire -, l'Ondam est au-dessous de l'inflation. Que les choses soient dites : en cette année de régression de l'épidémie, mais pas de fin de l'épidémie de covid-19, vous faites des économies sur le système de santé.

elles sont inférieures à l'inflation, dont je rappelle qu'elle est évaluée entre 6,2 % et 6,5 % cette année, et autour de 5 % en 2023. Certaines mesures sont positives, bien sûr, comme dans tout PLFSS.

Mais le texte ne prévoit rien pour répondre à l'urgence de l'affaissement de notre système hospitalier. Il ne comporte aucune réflexion sur l'Ondam, dont la construction doit être revue en profondeur. dépit des propos du ministre de la santé et de la prévention, le Gouvernement s'en tient à une stricte politique de l'offre, au lieu d'entamer la conversion vers une politique des besoins en santé du pays. Le rendez-vous avec la prévention reste ainsi largement esquivé.

fortement ? Nous nous réjouissons que ce soit le Sénat qui ait rétabli la version initiale du texte concernant le tabac à chauffer. Celle-ci n'est certes pas révolutionnaire, mais elle a le mérite d'avoir un impact. À l'avenir, il serait préférable que le ministre chargé des comptes publics évite de se rendre au congrès des buralistes avant de défendre le PLFSS dans cet hémicycle ... Nous avons le devoir de protéger la jeunesse.

interdits. Bien que notre amendement visant à aligner la fiscalité de l'alcool sur l'inflation n'ait pas été adopté, je me réjouis de l'avis courageux qu'il a reçu de la rapporteure générale et de la commission. De même, je salue l'adoption par le Sénat de la taxe sur les prémix à base de bière et de sucre. Ces votes sont d'autant plus importants que le Gouvernement n'a pas proposé grand-chose en la matière. Même constat sur la santé environnementale, dont les conséquences sur notre système de soins font pourtant

grand âge. C'est un renoncement. Devons-nous nous satisfaire de cette branche à déficit ? Le Gouvernement renonce-t-il à toute ambition forte en la matière ? Enfin, ce PLFSS a bien failli contenir une réforme des retraites. Celle-ci est en discussion et nous aurons bientôt, semble-t-il, l'occasion d'en débattre.

L'an dernier, j'avais dédié notre vote à l'hôpital public. Cette année, à cette tribune, c'est au personnel soignant que je le dédie. En 2020, les soignants étaient épuisés, mais fiers d'avoir accompli leur devoir face à la violente épidémie qui nous avait frappés. En 2022, ils sont épuisés et lassés des conditions de travail ou d'exercice qui se dégradent sans cesse. Ils sont au coeur d'un service public essentiel et précieux : nous leur confions l'état de santé de nos concitoyens. Madame, monsieur les ministres, vous entamez votre première année au sein de grands ministères. Je vous souhaite de porter les thématiques de santé publique, d'accès et de qualité des soins. soins. Démarquez-vous de cette logique comptable et de la mainmise de Bercy sur nos politiques de santé. À défaut, vos propos volontaires resteront des mots, et nos soignants, eux, renonceront de plus en plus. La parole

Après une semaine de débats, le bilan est toujours négatif, d'autant que la majorité sénatoriale l'a alourdi. Si nous nous réjouissons notamment de l'annulation du transfert à l'Urssaf du recouvrement des cotisations au de la suppression du transfert de charges de 2 milliards d'euros de la branche maladie à la branche famille et du rétablissement de la compensation des exonérations de cotisations de la prime de partage de la valeur, ces modifications ne permettent pas de revenir sur l'équilibre global du PLFSS pour 2023. Le Gouvernement prévoit une progression des dépenses de la branche assurance maladie de seulement 3,7 %, quand il faudrait que celle-ci soit de 4 % pour tenir compte uniquement de l'évolution naturelle des dépenses de santé. Chacune et chacun le sait ici : la hausse de 4,1 % du budget des hôpitaux demeure au-dessous du niveau de l'inflation, estimée par la Banque de France à 4,7 % pour 2023. Les affirmations d'autosatisfaction du ministre Attal n'y changent rien. C'est la première fois que l'Ondam est inférieur à l'inflation. C'est d'autant plus grave que certaines estimations prévoient une inflation à 6 %, ce qui revient à réaliser entre 1 et 2 milliards d'euros de coupes drastiques aux dépens de l'hôpital public. Ainsi, vous allez une fois encore réduire les dépenses des hôpitaux, ce qui va entraîner des fermetures de lits d'hospitalisation, de services et d'hôpitaux de proximité dans tous les territoires. Comment ne pas être en colère, révolté de constater que le groupe Les Républicains et le Gouvernement sont incapables de faire l'autocritique de l'échec des politiques de réduction des dépenses de santé ? Cela fait trente ans que notre système de santé est gangrené par votre logique libérale mortifère ! Nous en voyons les résultats des décennies de coupes budgétaires ont imposé un travail de plus en plus pénible à l'hôpital ; des organisations maltraitantes qui usent les personnels et dégradent la qualité des soins. Les personnels du secteur de la santé et du médico-social sont pourtant profondément attachés au service public et à la qualité de la prise en charge des patientes et des patients. Mais après une période aussi éreintante que la covid-19 et les sacrifices personnels du Gouvernement a fait déborder le vase. Désormais, même les plus convaincus du sens de l'intérêt général quittent le navire, parce qu'ils ont le sentiment d'être en contradiction avec leurs valeurs lorsque, faute de lits et de personnel suffisant, ils réalisent un tri des malades et laissent des heures entières des personnes âgées sur les brancards. Comme le souligne le collectif Inter-Hôpitaux dans une tribune publiée dans il y a quelques jours, « cette dégradation de la situation hospitalière risque d'aboutir à la disparition de pans entiers d'activités et de savoir-faire, dont l'hôpital public est le seul opérateur. La crise de la pédiatrie aujourd'hui préfigure ce qui arrivera demain pour l'ensemble de l'hôpital public ». Face à cette situation, le Gouvernement et la droite sénatoriale préfèrent maintenir les internes une année supplémentaire en stage dans des cabinets médicaux ou dans des hôpitaux pour cacher la misère, plutôt que de financer la santé à la hauteur des besoins. Cette situation n'est pourtant pas inexorable, et il n'est pas utopiste de trouver les 5 milliards d'euros nécessaires au recrutement de 100 000 professionnels et à la valorisation des métiers de l'hôpital. Le Gouvernement aurait pu décider, par exemple, de ne pas créer 5 milliards d'euros supplémentaires d'exonérations de cotisations sociales pour 2023, ou encore financer les 18 milliards de dépenses liées au covid-19 plutôt que de les faire peser sur le budget de la sécurité sociale. Cette volonté politique vous fait défaut, car elle va à l'encontre de votre projet politique de recul social. Si vous ne l'avez pas fait, c'est parce que vous voulez déstructurer l'hôpital public au profit du privé et fixer un panier de soins minimaliste au-delà duquel la prise en charge sera assurantielle. Tout au long de l'examen de ce PLFSS, nous avons pu constater un accord de fond entre le Gouvernement et la majorité sénatoriale : ils ont rejeté de concert tous nos amendements sur de nouvelles recettes, refusant notamment de supprimer les exonérations de cotisations patronales sur les bas salaires ou de revenir sur le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), qui pèse lourdement sur le budget de la sécurité sociale. La droite sénatoriale a même ajouté de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les médecins retraités qui continuent d'exercer. Surtout, vous avez adopté l'amendement n° 102 rectifié, visant à reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans et à allonger la durée de cotisation à 43 annuités. Infondée, injuste, une telle disposition va à l'encontre de l'aspiration des 70 % de Françaises et de Français qui défendent une retraite à 60 ans pour toutes et tous. Vous avez le mérite de la constance, mes chers collègues

derniers. Ce PLFSS pour 2023 est un rendez-vous manqué pour les personnels hospitaliers, qui attendaient des mesures en rupture avec les choix antérieurs afin d'améliorer leurs conditions de travail. C'est un rendez-vous manqué pour la médecine de ville, les centres de santé, les personnels des Ehpad, les aides à domicile

au bout des ruptures de stock. J'ai été alertée par l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament sur les risques de pénurie d'un antibiotique courant. Une telle pénurie frappe déjà les États-Unis. Or comme vous le savez bien, il peut y avoir un effet domino sur l'ensemble des antibiotiques. Quelles mesures allez-vous prendre à court, moyen et long termes pour combattre ce phénomène structurel ? Pourquoi refuser de tirer les enseignements de la crise de la covid-19 ? Pourquoi vous obstinez-vous à poursuivre et à amplifier les mêmes politiques, dont l'échec est patent ? Pour l'ensemble de ces raisons, les sénatrices et sénateurs du groupe communiste républicain citoyen et écologiste,

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, avant d'aborder ce PLFSS, son contenu, ses forces et ses faiblesses, je souhaite souligner sa forte portée symbolique. Je le dis sans réserve : la qualité de nos débats- sans être d'accord sur tout -, entre les groupes, mais aussi avec les ministres, honore la République. Sur le terrain, dans l'opinion et même dans la sphère médiatique, les éloges sur nos travaux fleurissent. Que d'autosatisfaction ! Entendez-vous les mêmes remarques que moi, mes chers collègues ? « Les débats au Sénat sont plus intéressants à suivre que ceux de l'Assemblée nationale. » « Vous travaillez bien, au Sénat. » « Heureusement qu'il y a le Sénat. » Ces remarques ne sont pas le fruit du hasard. Elles sont fondées, et même méritées. L'examen du PLFSS est l'occasion de souligner la place, le rôle et la responsabilité du Sénat au moment précis où le cocktail fait d'une majorité relative et de groupes extrémistes et populistes puissants fragilise l'Assemblée nationale.

Prenons ce bénéfice, chers collègues ! Les sénateurs ne se contentent pas, comme je l'ai parfois entendu de manière pernicieuse à l'époque, de rencontrer les maires comme les visiteurs médicaux rencontraient autrefois les médecins. Non, les sénateurs ne se contentent pas de faire des relations publiques auprès des élus pour assurer leur réélection. Bien sûr, les sénatrices et les sénateurs représentent les territoires et les collectivités territoriales, et, au premier rang, les hussards de la République que sont les maires. Mais ils sont mieux que cela des législateurs à part entière, qui font la loi animés par l'intérêt général et le bien commun. Pour preuve, si certains regardent parfois de l'autre côté de l'Atlantique pour justifier une modification de notre Constitution, nous, sénateurs, nous ne devons pas regarder vers les

Vous donnez la priorité au « vieillir à domicile ». Le virage domiciliaire est une priorité et nous le soutenons. Mais, en l'espèce, les moyens d'accompagnement tels que l'APA ne sont plus soutenables pour les départements.

au volet familial. Le refus par le Gouvernement de revaloriser de moitié l'allocation de soutien familial en faveur des parents isolés est l'une des rares lueurs de ce PLFSS

telle mesure démontre le manque d'ambition du Gouvernement en matière de politique familiale et le refus de revenir à l'universalité des allocations familiales, qui passe par la suppression de leur modulation. Pour nous, la politique familiale n'est pas une politique sociale : c'est bien une politique familiale. Il convient d'ailleurs de s'atteler à la création de places de crèches- nous en avons discuté, monsieur le ministre. C'est une attente des familles, mais aussi une mesure indispensable pour assurer l'égalité hommes-femmes et accroître l'employabilité.

Nous sommes les défenseurs du dialogue social, non par dogmatisme, mais parce que les retraites Agirc-Arrco sont bien gérées par les partenaires sociaux. La seconde mesure, importante, est celle qui porte sur les retraites. Elle démontre notre volonté de préserver le modèle français redistributif en maîtrisant la part des redistributions sociales. sociales. Pour conclure, j'aborderai une question qui me tient à coeur. Notre système de santé est en train de craquer- je le dis haut et fort. Il souffre au moins autant du manque de moyens que de la suradministration ou de la surbureaucratisation, un mal bien français. Je prendrai un dernier exemple. Conscients de la pénurie de médecins que connaît notre pays, nous avons voté à l'unanimité la fin du.

sous peine de voir la pénurie de médecins d'aujourd'hui s'aggraver demain et après-demain. Le système est à ce point absurde que nos étudiants les plus brillants sont contraints de se rendre en Roumanie afin d'y être de leurs études. Comment comprendre qu'un grand pays comme la France serait moins capable que la Roumanie, ou d'autres pays, de faire évoluer, dans l'intérêt de tous, son système de formation ? Mes chers collègues, le groupe Union Centriste votera ce PLFSS, mais nous voulions, au travers de cette intervention, témoigner de la fragilité de notre système de santé et de l'urgence de débattre d'une grande loi Santé. La parole loi Santé. La parole est à M. Jean Louis Masson, pour la réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste d'aucun groupe.

groupe. Monsieur le président, madame, monsieur les ministres, mes chers collègues, notre système de santé est très fragile et ce PLFSS, que nous votons aujourd'hui, en est l'illustration.

Pourtant, chacun s'accorde à reconnaître que la prévention serait la réponse la plus adaptée aux maux dont souffrent les finances de la sécurité sociale. Certes, nous saluons la réduction du déficit, convaincus que la maladie de la dette n'a pas un bon pronostic. Cependant, ce PLFSS relève davantage d'une compression exercée afin de contenir une hémorragie que d'une prise en charge globale de la maladie.

Nous attendons avec impatience la tenue d'une conférence nationale des générations et de l'autonomie, qui doit réunir les acteurs de la politique de soutien à l'autonomie, avec une mission prospective de documentation des données démographiques, médicales et socioéconomiques du vieillissement et de la dépendance.

Le groupe RDSE n'a pas voté l'amendement de notre collègue René-Paul Savary, relatif au recul des droits à la retraite. Les partenaires sociaux se sont enfin réunis autour de la table ; ce serait leur envoyer un mauvais signal. Faisons-leur confiance Le président Emmanuel Macron a mis cette réforme à l'ordre du jour. Le groupe RDSE est conscient de la nécessité de réformer notre système de retraite. Nous espérons que cela se fera au moyen d'un accord avec les partenaires sociaux dans le cadre du projet de loi attendu en 2023.

Dans dix ans, les pratiques auront évolué sous les effets de l'intelligence artificielle et de la robotique. Les transferts de tâches seront nécessaires pour redonner du temps d'analyse et de synthèse aux généralistes. La quatrième année du troisième cycle des études de médecine générale, destinée à former aux pratiques médicales de terrain, est nécessaire. Sa finalité ne doit pas être l'envoi de médecins débutants afin de peupler les déserts médicaux. Il s'agit avant tout d'une année de formation dédiée à la spécialité de médecine générale, comme il en existe pour toutes les autres spécialités. Elle engendrera naturellement du temps médical dans les déserts médicaux.

Les futurs médecins doivent échapper au conventionnement sélectif punitif. Il est sage de laisser émerger, des discussions conventionnelles, des solutions consensuelles afin de repeupler les déserts médicaux, grâce à des temps dédiés dans les zones sous-denses, mais proposés à l'ensemble des praticiens.

Il en est de même des réseaux de santé, comme les secteurs de l'optique et dentaire pour l'instant. C'est une perte de liberté des professionnels et des patients. Notre collègue Alain Milon l'a très bien expliqué : avec les complémentaires santé n'existent ni de participation selon ses moyens ni de prestations selon ses besoins. Il faut s'interroger, sans tabou, sur une sécurité sociale universelle plus juste et moins coûteuse, et les complémentaires doivent devenir des supplémentaires.

Enfin, je poursuis mon combat pour une évolution vers un équilibre entre la part Beveridge et le système bismarckien de sécurité sociale : que la vieillesse et les accidents du travail et

Emmanuel Macron avait engagé ce mouvement au début de son précédent mandat ; nous encourageons le Gouvernement à aller plus loin. Malgré quelques avancées intéressantes et l'adoption de nos amendements, notre groupe se partagera équitablement entre abstentions et votes contre

au terme de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, force est de constater que, vingt-six ans après la première édition de ce texte, le contrôle démocratique des finances sociales- et des 600 milliards d'euros de dépenses publiques qu'elles représentent -reste un chantier en cours. La loi organique du 14 mars dernier avait pour objectif d'y contribuer, mais ses apports sont limités. Certes, pour la première fois, nous avons obtenu le montant des dotations des agences sanitaires financées par l'assurance maladie. Faut-il rappeler cependant que nous en disposions de manière détaillée, lorsque ces mêmes agences étaient financées par le budget de l'État ? Pour la première fois également, nous avons obtenu, quelques heures avant le vote sur l'article qui lui est consacré, le montant des différents sous-objectifs de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, l'Ondam, au million d'euros près. Pas plus cependant. Avec un montant de quelque 240 milliards d'euros, l'Ondam ne peut pas rester plus longtemps une telle boîte noire. C'est ce que nous avons voulu manifester en le rejetant, tout en précisant, dans le texte, les conditions dans lesquelles le Gouvernement devrait revenir devant le Parlement en cas de dérapage. Nous sommes un peu las de devoir quémander des chiffres qui nous sont pourtant dus. Une fois ce PLFSS voté, je vous demande donc, madame, monsieur les ministres, d'engager avec nous un travail très opérationnel sur la mise en oeuvre, pour le moins parcellaire, de la loi organique, organique, s'agissant des informations qui nous sont communiquées. Deuxième chantier d'importance, le financement de la sécurité sociale n'a pas davantage gagné en clarté cette année. La commission conteste, chaque année, le calibrage du transfert de la branche des accidents du travail au titre de la sous-déclaration. De la même manière, si l'on peut comprendre l'intérêt de ne pas creuser durablement les déficits d'une branche, alors que d'autres sont en excédent, comment concevoir de faire porter à la branche famille 60 % du coût des congés maternité, alors que les indemnités journalières resteront bien versées, en totalité, par la branche maladie ? Avec cette mesure, on touche à une forme de raffinement technocratique qui caractérise parfois ce texte, mais qui confine, dans le cas d'espèce, à l'absurdité. Le congé post-accouchement n'est pas plus que la grossesse un mode de garde, mais il relève bien de la santé ! Par conséquent, nous avons rejeté ce transfert. Cette année encore, nous n'avons pas échappé à des débats de fiscalité sectorielle. À titre personnel, je suis favorable au transfert à l'État de cet inventaire à la Prévert de taxations diverses n'ayant qu'un lointain rapport avec la protection sociale.

À force d'être illisible, le financement de la sécurité sociale pourrait en devenir illégitime aux yeux de nos concitoyens. Le financement des solidarités n'est pas l'affaire des seuls spécialistes. La place des complémentaires notamment, dont nous avons pérennisé la taxation, doit ainsi être clarifiée. Troisième chantier d'importance, l'avenir. Avant la crise sanitaire, la sécurité sociale peinait à retrouver l'équilibre. Pour ses deux principaux postes de dépenses, la maladie et la retraite, les déficits sont structurels. Ils tiennent pour une large part au vieillissement de la population. Une population qui vieillit voit croître ses besoins en transferts sociaux, tandis que les générations les plus jeunes sont moins nombreuses pour les financer et sont confrontées à leurs propres besoins. Nous sommes fiers de notre modèle solidaire de protection sociale et nous avons raison. Cependant, la démographie le met singulièrement à l'épreuve, au risque, si nous ne faisons rien, de sa remise en cause. Nous avons voulu apporter des réponses concrètes sur la démographie médicale, l'intérim, les biologistes ou encore les téléconsultations. Nous espérons qu'elles seront reprises, tout comme le régime social des rachats de jours de RTT ou la pérennisation du dispositif

la garantie que la solidarité nationale sera bien présente pour eux aussi. La pérennité de notre modèle social suppose de le réformer, de façon continue, pour l'adapter aux mutations de la société et à l'évolution de ses besoins. des retraites complémentaires Agirc-Arrco, le Sénat s'est aussi inquiété de la pérennité de ce modèle et a supprimé le recouvrement par l'Urssaf. À cet égard, même si je n'élude pas celle de l'emploi des seniors, la question des retraites peut finalement paraître assez simple, une affaire de paramètres ... Celle de la dépendance est, en revanche, devant nous. À l'horizon de quelques années, les besoins connaîtront une augmentation très importante et les conditions d'un accompagnement digne des plus âgés ne sont pas en place. Il nous manque en particulier toutes les phases intermédiaires entre le domicile et l'établissement, dont les bases sont à peine posées. Comment rendre solvables des personnes ayant besoin de l'accompagnement d'un tiers, tout en vivant elles-mêmes de revenus de transfert ? Notre commission avait proposé qu'une assurance se développe sans tarder, car la dépendance est bien un risque et non une fatalité. Ce sera l'objet de la conférence nationale des générations et de l'autonomie, que nous avons souhaité instituer. Ces différents constats de carence nous ont conduits à rejeter la trajectoire proposée par l'annexe B, qui ne dessine en rien une stratégie, bien qu'elle intègre une réforme des retraites, mais dont les paramètres sont inconnus. Permettez-moi, pour conclure, même si j'interviens au nom de mon groupe, de saluer une nouvelle fois le travail des rapporteurs de la commission, qui, malgré des conditions particulièrement dégradées, ont su nous proposer des axes structurants pour l'examen de ce texte. C'est grâce à leur travail que le groupe Les Républicains se prononcera en faveur de ce texte. La parole

Monsieur le président, madame, monsieur les ministres,

Les orientations que nous impulsons cette année répondent à de nombreux besoins de nos citoyens. Je salue le travail effectué, au sein de la commission des affaires sociales, par notre rapporteure générale et nos rapporteurs. Je me félicite de la richesse des échanges en séance publique. Alors que nous faisons encore face à des tensions dans de nombreux secteurs de la santé, je souhaite remercier l'ensemble des soignants pour leur engagement et leur travail quotidien au plus près des Français. Les soins et l'offre de soins sont essentiels et doivent être répartis sur l'ensemble du territoire afin que chacun puisse en bénéficier. C'est notre objectif absolu. Il en est de même de la prévention, point sur lequel j'aimerais particulièrement revenir. Je pense Je pense que nous devons poursuivre nos efforts dans ce domaine. L'information des Français, la formation des professionnels et les dépistages permettent d'éviter des situations qui pourraient s'aggraver rapidement. Les trois consultations préventives à des âges clés de la vie sont un bon moyen de répondre à cet objectif. La prévention est essentielle pour la protection de nos enfants ; j'y suis très attachée. Il faut la développer afin de lutter contre les différentes formes d'addictions auxquelles les jeunes sont confrontés. Les tiers-lieux sont d'ailleurs une piste intéressante afin d'approcher certaines personnes en milieu rural ou dans des quartiers des villes. de l'occasion de parler de prévention pour évoquer celle de la perte d'autonomie. Nous avons entendu les promesses faites et les évolutions entérinées. Il faut se concentrer sur les emplois dans ce secteur : c'est indispensable. La dépendance progressera entre 2020 et 2030 : selon les prévisions, 200 000 personnes supplémentaires seront concernées. Mon collègue Daniel Chasseing a évoqué un objectif de 50 000 emplois dans ce secteur. Nous devons poursuivre nos efforts. Revenir sur la perte d'autonomie me permet de mettre en lumière les personnes accompagnantes. Les aidants sont précieux et consacrent une grande partie de leur vie à l'aide d'un parent. Leur engagement, souvent source de sacrifices, doit être salué. Je me félicite donc de l'adoption de l'amendement concernant l'ouverture

L'ouverture de la prescription et de l'administration des vaccins à davantage de personnels de santé, comme les pharmaciens, les infirmières ou encore les sages-femmes, est une bonne chose. Concernant les pharmaciens, et plus largement le sujet des médicaments, je me félicite de l'adoption de l'amendement ayant trait à la sécurisation de la filière de la vente en gros de médicaments : sujet ô combien crucial d'octobre, j'ai alerté le Gouvernement sur l'existence d'une pénurie des médicaments en France. Les tensions sur certains médicaments- les antidiabétiques, les anticancéreux ou encore ceux qui luttent contre l'hypertension -ne doivent pas persister. Une réorganisation structurelle, comme évoquée par le ministre, est nécessaire. Notre groupe est très engagé sur ce sujet. Autres avancées notables : la pilule du lendemain, gratuite pour toutes les femmes, sans ordonnance, ou encore le dépistage des infections sexuellement transmissibles, afin d'éviter leur propagation,

Je sais le bruit et les oppositions que ce sujet provoque. La rémunération, versée lors de cette année supplémentaire, est prévue par voie réglementaire. Elle doit être suffisante. Ce sujet me permet d'aborder celui des déserts médicaux. L'article voté ne suffira malheureusement pas à résoudre le problème. L'offre de formation doit aussi être

Ce genre de pratique doit faire partie du panel des solutions envisagées afin de lutter contre le manque d'offre de soins et de personnels soignants au sein de nos territoires. Le second sujet en suspens est celui de la téléconsultation,

Ce sujet est passionnant pour l'évolution de la médecine : nous allons au-devant d'innovations qui nous permettront de progresser encore davantage. Attention cependant, tout ne peut pas se faire en télémédecine. l'importante réforme des retraites. Le travail est en cours et nous attendons l'arrivée rapide d'un texte ; nous espérons une proposition de réforme dans les prochaines semaines. Si cela n'était pas le cas, notre groupe prendrait ses responsabilités. L'avenir des Français en dépend. de financement de la sécurité sociale marque des avancées importantes, même si de nombreux points restent en suspens. Malgré tout, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte.

ce premier PLFSS du deuxième quinquennat aurait dû enfin tracer les lignes d'une stratégie ambitieuse et au long cours, tenant compte des enseignements de la crise sanitaire, en faveur d'une politique sociale et sanitaire à la hauteur des enjeux. Tel n'est toujours pas le cas et nous ne pouvons que déplorer votre impéritie. Avant la pandémie, en 2019, des milliers de chefs de service vous alertaient et menaçaient de quitter l'hôpital en raison de l'incapacité de garantir des services de qualité.

Oui, du tri ! En 2022, en France, alors que l'épidémie est comparable à celle de 2012. Cependant, depuis cette date, l'hôpital public a continué de s'effondrer. Or lui seul assure la pédiatrie. Ce qui est un scandale, monsieur le ministre, ce n'est pas que les soignants parlent de tri, c'est de les obliger à en faire ! Qu'avez-vous fait pour la pédiatrie depuis cinq ans ? Le Gouvernement refuse de fixer un Ondam à la hauteur des enjeux, mais il débloque 400 millions pour passer l'hiver quand le scandale enfin éclate : cela ne fait pas une politique de santé. Cette gestion nourrira les démissions, une fois l'urgence passée. Nous le réaffirmons, seule une vraie perspective pluriannuelle peut donner du sens au nouvel effort que vous demandez au personnel hospitalier épuisé. Vous avez fermé des lits, supprimé des postes, planifié une gestion du personnel fondée sur des heures supplémentaires et des primes plutôt que sur des embauches et des revalorisations pérennes, et provoqué souffrance au travail, départs et suicides. Comme en matière d'inaction climatique, vous faites l'objet d'une action en justice à faire reconnaître la responsabilité de l'État dans la situation de l'hôpital public. Nous trouvons indécente la satisfaction du ministre des comptes publics s'agissant du niveau de l'Ondam. Votre aveuglement devient dangereux.

Vous préférerez systématiquement le calcul comptable aux défis sanitaire et social. Ainsi, vous multipliez les mesures d'exonération de cotisations sociales, dont la part non compensée est en hausse. La Commission des comptes de la sécurité sociale note ainsi que « les crédits affectés par l'État au titre de la compensation des exonérations seraient inférieurs de 4,3 milliards au coût global des mesures sur 2022 ». Ces milliards volés au budget de la sécurité sociale représentent plus de dix fois

Oserez-vous y revenir par un prochain 49.3, au mépris des deux chambres ? De manière générale, la trajectoire financière présentée a fait l'objet de nombreuses critiques. Elle trace l'horizon de pressions sur les dépenses publiques, notamment sur les retraites. Sur ce dernier point, nous devons marquer, une fois encore, notre opposition à la disposition introduite pour reculer l'âge de départ, là aussi avec les mêmes points aveugles sur la question des recettes, sur les politiques d'intensification du travail, de pénibilité et d'éviction des salariés les plus âgés, insuffisamment productifs et trop coûteux pour le capital, car, si la moitié des seniors sont hors de l'emploi au moment de la retraite, 47 % le sont pour cause de licenciement. À l'insuffisance de l'Ondam répondent les maigres ressources allouées à la branche autonomie. Nous ne reviendrons pas sur le coupable retard pris dans la prévention de la perte d'autonomie. Les mesures qui y sont attachées ne provoqueront pas le nécessaire choc d'attractivité, qui permettrait d'ouvrir enfin les 93 000 postes supplémentaires d'ici à deux ans pour les seuls Ehpad et autant pour pour le soutien à domicile associatif, qui attend les mesures spécifiques du Ségur pour mettre fin à un sous-effectif alarmant. Sur les autres enjeux, le texte se montre aussi insuffisant : alors que plus de 3 millions de personnes vivent dans un désert médical, le Gouvernement refuse d'envisager les premières mesures structurelles à même de desserrer la pénurie à court terme. La quatrième année d'internat ne peut être au service de la régulation, elle ne peut se justifier que pour la professionnalisation. D'autres pistes restent inexplorées. mondiale de la santé (OMS) montrent qu'il faut mettre l'accent sur la diversité sociale et géographique des étudiants en médecine, en favorisant l'inscription d'étudiants originaires de zones sous-denses, notamment rurales, et en déconcentrant l'enseignement. ce que nous avons proposé, en vain. Si le Gouvernement régule enfin la télémédecine, il ne peut s'empêcher un nouvel effet de loupe sur les arrêts maladie. Nous approuvons la suppression par le Sénat du transfert de charges de la branche maladie vers la branche famille. D'autant que nous avons souligné le caractère restrictif des mesures présentées en faveur de la famille, limitées aux familles monoparentales. De fait, le texte oublie certains foyers modestes. Rappelons que la pauvreté touche un enfant sur cinq. Il faut affecter une partie des excédents pour rouvrir les embauches nécessaires à la Cnaf, revaloriser le congé parental pour en faire non plus une trappe aux femmes pauvres, mais un choix partagé par les deux parents. Pour le moment, quatre enfants sur dix ne bénéficient pas d'un mode d'accueil. Si nous pouvons saluer la prolongation jusqu'à 12 ans du complément de libre choix du mode de garde (CMG), ainsi que les dispositions pour prévenir la récidive des impayés des assistantes maternelles, il reste que nous manquons ici l'occasion de relancer une politique au profit des familles et des femmes. Car, à la source des inégalités entre les femmes et les hommes, on trouve souvent des carrières interrompues, des temps partiels subis pour s'occuper d'enfants à qui aucun autre mode de garde n'est offert. en soulignant que ce PLFSS pour 2023 sonne de nouveau comme un rendez-vous manqué. Ce manque de vision stratégique, au moment où l'hôpital public traverse crise sur crise et alors que la lutte contre la pauvreté marque le pas, explique le vote contre du groupe Écologiste- Solidarité et Territoires. Il va être et Territoires. Il va être procédé, dans les conditions prévues par l'article 56 du règlement, au scrutin public solennel sur l'ensemble du projet de loi, de financement de la sécurité sociale pour 2023.

tout d'abord, je souhaite remercier la Haute Assemblée pour la qualité des débats que nous avons eus, sur les branches autonomie et famille en particulier. Je salue l'esprit constructif de la rapporteure générale, Élisabeth Doineau, et des rapporteurs Philippe Mouiller et Olivier Henno, avec lesquels le dialogue a été, dès le premier jour, franc, ouvert et constructif. Au-delà, j'ai été heureux de constater l'engagement, sur ces sujets si importants, de l'enfance au grand âge, en passant par le handicap, Le texte qui vous avait été présenté était, dès le départ, très ambitieux : 1,5 milliard d'euros supplémentaires pour la branche autonomie et 1,6 milliard pour la branche famille. Il a été progressivement enrichi à l'Assemblée nationale puis ici.

loi. Je retiens surtout une véritable convergence de vues sur les grands enjeux. D'une part, garantir à nos aînés des conditions de vie à domicile ou en établissement dignes, sécurisantes, avec le soutien de professionnels en nombre suffisant. D'autre part, adapter les outils de notre politique familiale aux besoins et aux attentes des familles, avec une attention particulière pour les plus fragiles, les familles monoparentales.

Il symbolise le dialogue de qualité que nous avons su construire avec l'Assemblée des départements de France, dont je salue de nouveau son président, François Sauvadet. Je sais que les questions relatives à la situation financière des établissements et services du grand âge ont aussi retenu votre attention. attention. À ce titre, je suis très heureux de vous signaler la publication, hier, du décret sur le bouclier tarifaire, dans lequel figurent bien les Ehpad. Je salue d'ailleurs la sénatrice Laurence Muller-Bronn, avec laquelle nous avions eu l'occasion de travailler sur ce sujet dès cet été. de la branche famille, je ne doute pas que vous serez nombreux à suivre avec attention, ces prochaines années, le déploiement des grandes réformes engagées par le Gouvernement. Je tiens à signaler en particulier celle qui porte sur le complément de libre choix du mode de garde, structurante et directement utile à de nombreux foyers, mais également la création du service public de la petite enfance- et je sais que vous serez particulièrement attentifs à ce que les collectivités conclure, je veux saluer de nouveau, comme je l'ai fait dès le premier jour des débats, l'action de tous les professionnels du soin, de tous les professionnels du lien, dont nous reconnaissons tous le rôle décisif. Ce texte est également pour eux, puisqu'il finance par exemple la trajectoire de recrutement de 50 000 professionnels supplémentaires dans le secteur médico-social, en Ehpad, au cours des prochaines années.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure générale, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, tout d'abord, je vous prie d'excuser l'absence de François Braun, retenu à l'Assemblée nationale par la séance de questions au Gouvernement.

qu'en 2017, avec un budget de 244 milliards pour la partie santé ! Je tiens à le souligner, ce projet de loi, c'est d'abord celui de la défense de l'hôpital : pour la deuxième année consécutive, aucune économie ne lui est demandée.

Il prévoit aussi des mesures concrètes pour lutter contre les déserts médicaux et pour avancer vers la société du bien vieillir chez soi. Le Sénat a porté des exigences fortes pour favoriser la transparence dans les Ehpad et renforcer nos dispositifs de lutte contre les fraudes. Nous avons pu diverger sur les moyens, mais le Gouvernement partage pleinement ces ambitions. ma conviction est que ce PLFSS porte une ligne claire, celle de la défense des préoccupations essentielles de nos concitoyens : plus de prévention, un accès renforcé aux soins, un système plus juste et plus éthique. C'est une première pierre de la politique de refondation que nous voulons engager avec la volonté- c'est notre horizon -de répondre à tous les besoins de santé de tous nos concitoyens. Je souhaite remercier

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

il y a deux ans, nous avions adopté une résolution pour la paix en Arménie et pour condamner l'agression contre le Haut-Karabagh commise par les

Bien sûr, une mission d'observation a été dépêchée, mais le temps n'est plus à observer : il est désormais à décider ; le temps n'est plus à protester : il est à sanctionner, et c'est précisément ce que nous proposons par cette résolution,

une forme de relativisme de la part d'une Europe oublieuse de ses valeurs, de ses principes, oublieuse aussi de ses propres racines. Mes chers collègues, si ce sentiment de honte nous est étranger, alors peut-être qu'un sentiment de crainte, de peur, pourrait nous saisir. Quel est-il,

ce conflit n'est pas un conflit local : il s'inscrit dans une stratégie turque globale visant à reconstituer un grand ensemble néo-ottoman, un ensemble

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cette proposition de résolution a une première vertu, que vient d'ailleurs de rappeler le président Retailleau outre la possibilité qui nous est offerte ici de débattre et de réaffirmer les positions qui sont les nôtres pour aller vers une paix durable, elle nous permet d'apporter un soutien sans faille aux peuples en souffrance, aux peuples qui ploient sous le joug de la guerre et du nationalisme. Nous n'exprimerons jamais assez notre totale solidarité à la population arménienne, comme le font depuis toujours les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, population victime du conflit de 2020, qui a fait plus de 6 500 morts,

Ce peuple qui a tant souffert doit voir revenir tous les éloignés dans leurs foyers : nous appelons à la libération et au rapatriement immédiats et inconditionnels de tous les prisonniers de guerre arméniens. Du territoire de l'Arménie et du couloir de Latchin, nous demandons le retrait immédiat et inconditionnel, sur leurs positions initiales, des forces azéries et de leurs alliés. Les autorités azéries et l'ensemble de leurs partenaires dans la région doivent respecter l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Arménie. Les engagements internationaux existent : ils doivent être suivis d'effet. À l'évidence, le cadre de sécurité dans lequel est entrée l'Arménie depuis le cessez-le-feu lui assure un faux-semblant de sécurité : il n'a échappé à personne que l'Azerbaïdjan a tenté de maximiser ses gains territoriaux.

Pour autant, il convient de rester attentif. Ce conflit ne peut être l'otage de l'instabilité dans le Caucase et des stratégies développées par les grandes puissances régionales. Nous l'avons constaté : la médiation russe de la force d'interposition de l'Organisation du traité de la sécurité collective (OTSC) n'est plus en mesure de stabiliser le conflit à moyen ou à long terme. la France, au sein de l'Union européenne, doit jouer son rôle. Le Président de la République a évolué sur ce dossier : tant mieux. Mais il doit bouger encore plus vite, et l'Europe avec lui. L'Union européenne doit adopter sa propre stratégie à propos du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, en soumettant les achats de gaz à l'Azerbaïdjan au respect du droit international. Le Gouvernement doit amplifier ses initiatives permettant de garantir la sécurité des populations arméniennes et de l'Arménie, dans ses frontières internationalement reconnues.

À plus long terme, l'Union européenne doit inclure le conflit arménien dans le cadre de la gestion des tensions régionales, dans un périmètre plus large. Les déflagrations de cette région, qui s'étendent de l'Europe orientale à l'Asie centrale, sont susceptibles d'avoir des répercussions sur des États voisins de l'Union européenne qui lui sont ou lui seront liés un jour par des partenariats. Mes chers collègues, en défendant cette proposition de résolution, nous manifestons notre soutien à un règlement pacifique du conflit, au maintien des principes de la démocratie et de l'État de droit chez les deux

Il est temps de revenir à la raison et de retrouver la voie du dialogue. Il est temps de satisfaire l'Arménie et les Arméniens dans leur volonté d'une paix juste. Il est temps d'aboutir, enfin, à l'établissement d'une paix durable dans cette région du monde.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en septembre dernier, une délégation du Sénat a été reçue à Erevan par les autorités arméniennes notre collègue et ami le député Vladimir Vardanyan, président du groupe d'amitié Arménie-France, nous a dit, les larmes aux yeux, sa terreur de ne pouvoir éviter à son peuple un second génocide. En octobre 2019, nous étions tous les deux dans la clairière du Mont-Valérien, là même où Missak Manouchian fut fusillé par les Allemands le 21 février 1944. Missak Manouchian a donné sa vie pour la liberté de la France. Que sommes-nous prêts à donner à l'Arménie pour sa liberté ? Du 27 septembre au 10 novembre 2020, la République d'Artsakh a subi l'invasion militaire de l'Azerbaïdjan, aidé par la Turquie et renforcé par des groupes djihadistes venant de Libye et de Syrie. La Turquie a ainsi participé, au moins indirectement, à un conflit de haute intensité selon une doctrine et des processus militaires qu'elle a appris au sein de Ce sont les mêmes tactiques que l'Ukraine utilise aujourd'hui avec succès contre l'invasion russe. Ainsi, les drones turcs Bayraktar TB2, employés par l'Ukraine, sont également mobilisés par l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Israël fournit aussi des drones aux deux armées. La République d'Artsakh et l'Arménie ont été totalement dépassées par l'ampleur et la violence de ce conflit d'un nouveau genre. Elles n'ont dû leur survie qu'à la mansuétude de la Russie, qui voulait démontrer, en 2020, que la sécurité du Caucase ne dépendait que d'elle. C'est sans aucun doute le désastre militaire de l'armée russe en Ukraine qui pousse aujourd'hui l'Azerbaïdjan à profiter de son avantage pour imposer par la force à l'Arménie un redécoupage des frontières internationales à son profit. Son objectif stratégique est connu. Il consiste à établir une continuité territoriale avec sa République autonome exclavée du Nakhitchevan en annexant un corridor le long de la frontière entre l'Arménie et l'Iran. Cette ambition n'est qu'une déclinaison régionale du grand projet panturquiste de constitution d'un espace politique unifié d'Istanbul à Bichkek, au Kirghizistan. En octobre dernier, la France, par la voix de son Président, a explicitement caractérisé les agressions de l'Azerbaïdjan comme une violation des frontières arméniennes reconnues par le droit international. Il est affligeant qu'en juillet la présidente de la Commission européenne se soit rendue à Bakou pour sceller un accord énergétique avec l'Azerbaïdjan, ... C'est une honte ! ... qualifié de partenaire de confiance. Scandaleux ! L'Azerbaïdjan exporte plus de pétrole qu'il n'en produit et vend sans doute à l'Europe une partie du pétrole qu'il reçoit de la Russie. pays s'est aussi engagé à doubler ses exportations de gaz vers l'Europe ; or le principal champ gazier azéri est notamment exploité par la compagnie russe Lukoil. Nous sommes prêts à oublier tous nos principes moraux quand il s'agit d'assurer la sécurité des approvisionnements énergétiques de l'Europe et singulièrement ceux de l'Allemagne. Depuis plus d'un siècle, l'Arménie est le miroir de nos lâchetés, de nos hypocrisies et de nos trahisons. Très bien ! Aussi, nous sommes très favorables à cette proposition de résolution, qui demande notamment au Gouvernement de mobiliser sa diplomatie pour obtenir de l'Union européenne un embargo sur le pétrole et le gaz provenant d'Azerbaïdjan. Mais, au-delà, comment assurer durablement la survie de l'Arménie ? De nombreux Arméniens pensent trouver leur sécurité sous la tutelle russe et le catholicos de l'Église apostolique arménienne vient de recevoir de Vladimir Poutine les insignes de l'ordre de l'Honneur. Le soutien de la Russie s'est déjà révélé défaillant par le passé. Aujourd'hui, son intérêt stratégique est de prolonger ce conflit pour maintenir l'Arménie dans un état de subordination et faire valoir cette protection relative dans une négociation plus ample. De nouveau, les conflits ukrainien et arménien sont liés. Pour aider durablement l'Arménie, il revient à la France et à l'Europe de poser les bases d'un nouveau multilatéralisme à l'échelle du continent européen et de son proche environnement. Cette réflexion ne peut éluder les problèmes posés par nos relations avec la Turquie et ceux de son projet expansionniste. Son appartenance à l'Otan ne justifie pas l'abdication collective de l'Europe face à l'agression turque contre l'Arménie. Elle ne justifie pas davantage les manoeuvres de la Turquie contre la Grèce et l'occupation militaire d'une partie du territoire de la République de Chypre. Avant d'être fusillé, Missak Manouchian écrivait à sa femme : « Je suis sûr que le peuple français et tous les combattants de la liberté sauront honorer notre mémoire dignement. » Aujourd'hui, le peuple arménien nous demande de rester fidèles aux combats de la France pour la liberté et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La

l'Azerbaïdjan. Plus de 6 500 personnes ont alors été tuées. Les armes se sont tues à la suite d'un cessez-le-feu publié le 10 novembre 2020. Des affrontements sporadiques ont eu lieu au cours de l'année 2021. Plus récemment, dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier, le cessez-le-feu a de nouveau été rompu. L'Azerbaïdjan a envoyé des troupes sur le territoire arménien, où elles se sont installées : il s'agissait, selon Bakou, d'une réponse à des provocations arméniennes. Le bilan est tout de même de 286 morts et, malheureusement, ces affrontements de septembre- les plus violents depuis 2020 -ne s'apparentent pas à des incidents isolés. La semaine dernière, les deux pays se sont encore accusés mutuellement de bombardements frontaliers. frontaliers. Au nom du groupe Union Centriste, je condamne le recours à la force, qui ne peut être un outil de résolution des différends entre États. C'est tout particulièrement vrai lorsqu'ils appartiennent aux mêmes instances internationales, comme l'Arménie et l'Azerbaïdjan, membres du Conseil de l'Europe, du Partenariat oriental de l'Union européenne et, en vertu d'une adhésion plus récente, de la Communauté politique européenne. Pour retrouver le chemin de la paix, l'intégrité territoriale de l'Arménie doit être respectée et préservée. L'Azerbaïdjan doit donc se retirer du territoire arménien, conformément à l'accord de cessez-le-feu de novembre 2020 ainsi qu'à la déclaration d'Alma-Ata de 1991. Les deux États doivent respecter leurs engagements internationaux et s'atteler à négocier rapidement un accord de paix durable conforme à ces engagements, lequel devra bien sûr être respecté. Monsieur le ministre, le 6 octobre dernier, lors du sommet de Prague et de la première réunion de la Communauté politique européenne, un premier pas a été franchi en faveur d'un dialogue entre les deux États. A été décidé l'envoi d'une mission civile en Arménie, le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan, afin d'établir une confiance mutuelle entre les deux pays et de contribuer à la délimitation de frontières pérennes entre les deux belligérants. Quels sont les premiers retours de cette mission, placée sous l'égide de l'Union européenne ? européenne ? L'Union européenne veut jouer un rôle de médiateur dans le règlement de ce conflit. Elle est, en même temps, soumise à de forts enjeux stratégiques en matière d'autonomie énergétique : c'est la conséquence directe de la guerre en Ukraine et des sanctions imposées à la Russie. L'Union européenne a d'ailleurs signé cet été un nouveau partenariat énergétique avec l'Azerbaïdjan, renforçant ainsi ses relations bilatérales avec ce pays. Dès lors, comment être certain qu'elle pourra jouer son rôle d'arbitre sans être contrainte par d'éventuelles pressions ? ? J'attire également votre attention sur la préservation du patrimoine du Haut-Karabagh. Cette région constitue l'un des berceaux de l'humanité et elle est en péril. Dans un rapport relatif au Haut-Karabagh, dont je salue la qualité, notre assemblée alertait déjà en juillet 2021 quant au risque de destruction du « petit patrimoine », témoin de l'empreinte arménienne de la région. La communauté internationale et la France ne sauraient cautionner la politique de destruction du patrimoine culturel et religieux arménien, visant à effacer toute trace de la culture arménienne. Le Sénat s'est toujours tenu aux côtés de l'Arménie : en témoignent les différentes résolutions transpartisanes examinées dans cet hémicycle.

monsieur le ministre, chers collègues, face à l'agression scandaleuse dont l'Arménie est victime, l'inaction des États-Unis, de l'Union européenne et de la France a été et est tout à fait lamentable. C'est pourquoi la proposition de résolution qui nous est soumise est véritablement la bienvenue. Mais il ne faut pas seulement mettre en cause le dictateur Aliyev, qui préside l'Azerbaïdjan. Il faut aussi- et je dirais même surtout -mettre en cause le Turc Erdogan,

entendu, il n'a jamais accepté de reconnaître le génocide de 1915. Il ne l'a jamais désavoué et on peut même dire qu'il l'a approuvé.

on se dit : manifestement, la France ou tout au moins le gouvernement français cautionne ; l'Union européenne cautionne. On va rendre visite au dictateur d'Azerbaïdjan ; on le remercie

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le 9 novembre dernier, à Toulon, le Président de la République présentait la nouvelle revue stratégique nationale. Il soulignait à cette occasion : « L'agression contre l'Ukraine risque de préfigurer de plus vastes réalités géopolitiques à l'avenir, que nous n'avons nulle raison d'accepter avec fatalisme et que nous n'entendons pas subir avec passivité. Dans cet esprit, la proposition de résolution qui nous est présentée aujourd'hui nous invite à ne pas accepter la fatalité d'un conflit qui, s'il touche au premier chef l'Arménie et l'Azerbaïdjan, résulte également d'un jeu d'influence entre la Russie et la Turquie.

et d'une proximité culturelle qui ont toujours conduit la France à porter un regard des plus attentifs à la situation de ce pays. De la première guerre remportée en 1994 par les Arméniens à celle dite « des 44 jours », de l'automne 2020, gagnée cette fois-ci par l'Azerbaïdjan, le bilan humain est tragique. Les exactions commises, notamment, par les soldats azéris contre des Arméniens renvoient au douloureux souvenir du génocide arménien de 1915. Ces crimes ne devront pas rester impunis. En outre, ils ne devront certainement pas être documentés par Bakou, comme l'a demandé le porte-parole de la Commission européenne au sujet d'une vidéo mettant en scène des soldats violentés et assassinés. En septembre dernier,

Peut-être ; mais la réalité, c'est aussi que le Président Aliyev, fort d'une armée soutenue matériellement par la Turquie et alimentée par des drones israéliens, souhaitait depuis plusieurs mois voir de nouveau posée la question des frontières et celle du statut du Haut-Karabagh. Bakou, on s'est souvent enorgueilli des quatre résolutions adoptées par l'ONU en 1993, rappelant l'inviolabilité des frontières il faut le reconnaître -, les quatre rencontres organisées à Bruxelles depuis 2021, comme celle du 6 octobre dernier à Prague, lors du premier sommet de la Communauté politique européenne, ont échoué. Toutefois, il ne faut pas renoncer.

En revanche, gardons-nous de donner à cette guerre des ressorts religieux : une telle interprétation ne saurait traduire une réalité géographique complexe héritée d'une histoire ancienne. Il n'y a pas de croisade islamiste, mais il y a certainement des velléités de conquête ou de reconquête territoriale.

Toutes ces difficultés passées et présentes ne doivent pas décourager la communauté internationale ; nous devons garder notre objectif de paix dans cette zone du Caucase Sud, d'autant que l'Arménie se dit prête à avancer des propositions. Elle vient de le faire avec son projet de zone démilitarisée. Le RDSE soutient le Gouvernement et le chef de l'État dans leur recherche d'une issue diplomatique, que ce soit avec l'appui du Conseil de sécurité de l'ONU ou de l'Union européenne, le tout dans un souci d'équilibre entre les deux parties.

je tiens à saluer la diplomatie parlementaire. En 2020, sous l'égide de Gérard Larcher, de Bruno Retailleau et de tous les présidents de groupe de cette assemblée, nous avons voté la reconnaissance de l'Artsakh. les Arméniens ont dû de nouveau compter leurs morts, les corps mutilés par les bombes au phosphore et les bombes à fragmentation au Haut-Karabagh, lors d'une guerre asymétrique qui a fait tant de morts. Malgré nos alertes, malgré les votes des deux assemblées, malgré les cris des Arméniens, notre gouvernement a préféré la neutralité il prouve encore aujourd'hui sa passivité, comme l'a souligné le président Retailleau. Pendant la guerre des 44 jours, le ministre des affaires étrangères prônait la neutralité. Aujourd'hui, il semble indifférent à l'appel du Sénat.

tandis qu'à Bakou, le 10 décembre 2020, le président Erdogan rendait hommage à Enver Pacha, ministre de la Guerre en 1915 et architecte du génocide, en s'engageant à poursuivre son oeuvre ; comme si le drame des Arméniens devait encore se répéter. face à la passivité de la communauté internationale, pleinement mobilisée, à juste titre, par l'Ukraine, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, s'attaque non plus à l'Artsakh, mais à la République souveraine d'Arménie. personnes, soldats arméniens et civils, ont été massacrées en quelques heures, s'ajoutant aux plus de 6 500 morts déplorés lors de la guerre des 44 jours, en 2020. Les crimes de guerre sont fièrement exhibés sur la toile par des militaires azerbaïdjanais se filmant dans leurs oeuvres de viol, de torture et de démembrement. Toujours la même barbarie, toujours les mêmes crimes, toujours la même passivité des démocraties occidentales et, surtout, européennes : si l'histoire est un perpétuel recommencement, elle ne doit pas être un renoncement éternel. Ces crimes de guerre doivent être punis. Ne nous y trompons pas : nous sommes bien face à une nouvelle guerre de conquête aux portes de l'Europe. Bien sûr, depuis la chute de l'Union soviétique, se pose la question du statut de la région de l'Artsakh, territoire dont la majorité arménienne vit sous la menace permanente du nettoyage ethnique, des injures, des incursions et des opérations de terreur. Mais désormais s'y ajoute la question des frontières de la République d'Arménie. En effet, le président autocrate Ilham Aliyev ne se contente plus de massacrer les Arméniens de l'Artsakh : il attaque le territoire de l'Arménie, État reconnu par la communauté internationale. L'Institut Lemkin pour la prévention des génocides a d'ailleurs lancé, il y a un mois, sa troisième alerte en moins d'un an. Cette barbarie s'inscrit dans la logique génocidaire, bien présente dans le Caucase. N'oublions pas l'arménophobie et le racisme d'État pratiqué par l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie, lequel n'a pas vocation à s'arrêter aux frontières de ce pays. N'oublions pas que l'Europe aussi est menacée, notamment la Grèce et Chypre, occupée depuis 1974 par la Turquie. C'est précisément là qu'Aliyev et Erdogan ont fêté leur sombre victoire de 2020. de 2020. Ilham Aliyev a toujours déclaré vouloir chasser « ces chiens d'Arméniens », qu'Erdogan appelle quant à lui « les restes de l'épée », par allusion au génocide de 1915. Alors, demandons-nous pourquoi l'Europe, qui refuse à juste titre toute compromission avec la Russie dans la guerre en Ukraine, se contente d'être spectatrice de la guerre en Arménie. La vie des Arméniens vaut-elle moins que celle des Ukrainiens ? Rappelons-le : fin juillet, Aliyev a obtenu un blanc-seing de la Commission européenne sous la forme d'un accord gazier prévoyant le doublement des livraisons de gaz à l'Europe. Ursula von der Leyen voit d'ailleurs en Aliyev un « partenaire fiable et sur lequel on peut compter ». Quelle indécence ! J'invite la présidente de la Commission à se rendre, comme nous, sur les tombes de nos alliés arméniens

Comment a-t-on pu abandonner cette terre emblématique des chrétiens d'Orient, qui essaient d'y survivre au milieu d'un environnement hostile ? Au nom des valeurs qui sont les nôtres et pour lesquelles nous défendons l'Ukraine, il faut sauver l'Arménie. Notre tradition universaliste et humaniste de défense des droits de l'homme,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis un mois seulement, les canons se sont arrêtés. La rivalité entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan remonte à plus d'un siècle. En 1992 s'est constitué le groupe de Minsk afin de trouver par la négociation une solution politique au conflit.

Le multilatéralisme et la négociation politique sont incontournables pour aboutir à des avancées solides et résoudre définitivement ce conflit.

Notre pays doit oeuvrer à ce que l'Azerbaïdjan et l'Arménie reconnaissent mutuellement la souveraineté politique et géographique, ainsi que l'inviolabilité des frontières internationales de chacun, conformément à la Charte des Nations unies. C'est exactement l'objet de la réunion quadripartite entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la France et l'Union européenne qui s'est tenue le 7 octobre dernier à Prague. À cet égard, nous devons saluer l'initiative du président Macron. Cette rencontre a permis des avancées sur la délimitation des frontières entre les deux pays. Il a été convenu de mettre en place une mission civile de l'Union européenne le long de la frontière pour une durée de deux mois. Cette mission a commencé il y a une semaine. Il me paraît donc prématuré de prendre position avant d'en connaître les conclusions officielles. En attendant, En attendant, la France doit poursuivre son action afin de faire converger les points de vue, en toute neutralité et impartialité, comme elle l'a fait lucidement et discrètement entre Israël et le Liban- les deux pays, en guerre depuis quatre-vingts ans, ont récemment signé un accord historique sur la délimitation de leurs frontières. Ce n'est pas la position de tous les acteurs. À cet égard, le soutien de la Turquie à l'Azerbaïdjan, pour des raisons idéologiques et stratégiques, et son implication dans les agressions ne font que compliquer la situation, déjà conflictuelle. De même, il nous semble indispensable que le retour des populations déplacées par les combats et la libération des prisonniers de guerre puissent se faire en toute sécurité sous la supervision des Nations unies. À cet effet, nous demandons que les forces de maintien de la paix de l'ONU soient déployées tout le long de la frontière et dans les zones disputées, en remplacement des forces russes, qui ont échoué dans leur mission, convenue lors de l'accord de cessez-le-feu du 10 novembre 2020. Bien sûr, les auteurs des atrocités et des crimes de guerre doivent être jugés devant une juridiction internationale. La France et l'Union européenne doivent multiplier leurs pressions en ce sens, car, jusqu'à présent, ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan ne reconnaissent la Cour pénale internationale,

La culture arménienne est considérée comme l'une des plus anciennes au monde ; la société azerbaïdjanaise est multiethnique, multireligieuse et multiculturelle. Nous devons respecter l'identité de chaque peuple. La paix se construit dans l'acceptation de l'autre. Notre rôle est de promouvoir des valeurs de paix et de fraternité, qui permettront aux Arméniens et aux Azéris de renouer entre eux des relations qui n'existent malheureusement plus aujourd'hui. Nous devons éviter d'alimenter des haines en ouvrant la voie à la compréhension mutuelle.

Or le manque d'impartialité risque de compromettre notre position de médiateur et notre légitimité auprès de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. Je ne suis pas certain non plus que cela serve les intérêts du premier ministre Nikol Pachinian, car

qui ont fait 286 victimes. En outre, l'Azerbaïdjan devra vraisemblablement répondre devant les tribunaux internationaux de probables crimes de guerre commis contre les soldats arméniens. Une enquête internationale doit être diligentée sans délai pour qualifier ces exactions. Nous réitérons notre soutien inconditionnel au peuple arménien dont la nation, le territoire et la culture doivent impérativement être préservés. Le peuple arménien doit être garanti dans son droit à vivre en paix et en sécurité. Dans cette perspective, nous partageons les mots forts du Président de la République, qui a rappelé que la France ne lâcherait jamais l'Arménie. La reprise de ce conflit territorial, vieux de trois décennies, moins de deux ans après la fin de la guerre de 2020, est une nouvelle conséquence des déstabilisations géopolitiques provoquées par l'invasion russe en Ukraine. Ainsi, comme à leur habitude, l'Azerbaïdjan et la Turquie tentent, par tous les moyens, de profiter de la guerre en Europe pour pousser leurs avantages.

Tant que nous ne nous serons pas engagés massivement pour sortir des hydrocarbures, l'autonomie stratégique du continent demeurera une chimère. Pourtant, dans le contexte géopolitique actuel, fragilisée militairement et isolée diplomatiquement, ne peut demeurer le seul garant de la paix dans le Sud-Caucase. Il faut que la communauté internationale, par le biais des Nations unies plutôt que par celui du groupe de Minsk- dévitalisé -prenne les dispositions nécessaires pour garantir l'effectivité du cessez-le-feu et la construction d'une paix durable dans le Haut-Karabagh. Si la nécessité l'impose et si la cohabitation avec la force d'interposition russe est possible, alors il faudra déployer une force de maintien de la paix internationale sous égide onusienne. et c'est toute la difficulté de la période -d'envisager une quelconque intervention dans la région sans composer avec la Russie de Vladimir Poutine. Si une première médiation, entreprise par les États-Unis et l'Union européenne le 2 octobre dernier, a permis la libération de dix-sept prisonniers arméniens, c'est un sommet tripartite, organisé par la Russie, qui a débouché sur un engagement de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie « ne pas recourir à la force », avant que les États-Unis ne tentent de reprendre la main au moyen d'une réunion des ministres des affaires étrangères, le 7 novembre 2022. Cette construction d'un traité de paix, encore fragile, comme l'illustrent les échanges de tirs la semaine dernière, qui plus est, dans un contexte international extrêmement troublé, doit être encouragée par tous les moyens. La pacification de la région est une nécessité vitale pour l'Arménie, qui ne paraît pas en mesure de faire face à un regain des tensions militaires. Cela étant, si le groupe écologiste partage de nombreuses demandes de la présente proposition, il ne juge pas opportun d'inviter le gouvernement français à renforcer « les capacités de défense de l'Arménie Il juge même paradoxal de faire figurer une telle demande dans une résolution « visant à établir une paix durable ». Comment la France, membre du groupe de Minsk, pourrait-elle jouer un quelconque rôle de médiateur dans la région, si elle devenait ainsi partie prenante au conflit ? un rôle moteur- ce que nous appelons de nos voeux sur toutes les travées -, pour que la communauté internationale tout entière garantisse la paix dans le Sud-Caucase- et ainsi la préservation de la République d'Arménie -, alors elle ne peut pas jouer une autre partition que celle de la diplomatie.

avec le rôle que doit jouer la France dans l'effort de construction d'une paix durable, seule à même de protéger durablement et effectivement l'Arménie et son peuple. La

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le conflit qui oppose la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan s'inscrit dans la durée, puisque plusieurs épisodes de violences ont eu lieu depuis la proclamation de l'indépendance du Haut-Karabagh en 1991. La présente proposition de résolution vise, à son alinéa 17, à pousser le Gouvernement à agir pour faire respecter le cessez-le-feu du 9 novembre 2020.

Le Président de la République a eu samedi dernier un échange téléphonique avec son homologue azerbaïdjanais, à l'issue duquel les deux dirigeants ont souhaité « maintenir une étroite coordination ». Il s'entretiendra également avec le premier ministre arménien en marge du sommet de la francophonie à Djerba le 19 novembre prochain. La voie du dialogue permet d'avancer de façon concrète avec les deux parties. Il faut rappeler cette échéance et privilégier le dialogue entre dirigeants. La France souhaite s'inscrire dans une position de conciliation des intérêts et permettre le dialogue constructif entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. à Washington, le lundi 7 novembre dernier, sous l'égide des États-Unis, quelques heures après de nouveaux bombardements frontaliers, dans un conflit qui a fait des centaines de morts ces derniers mois. La France a « souhaité maintenir une étroite coordination dans le sillage du sommet de Prague », qui avait réuni le 6 octobre dernier, en marge de la première réunion de la Communauté politique européenne, le président Aliyev et le premier ministre Pachinian. Le Président de la République a « salué l'effet stabilisateur de la mission civile de l'Union européenne le long de la frontière avec l'Azerbaïdjan ». Le déploiement de cette mission avait été décidé lors du sommet de Prague. Le Président de la République a également réaffirmé « la pleine disposition de la France à accompagner le processus de normalisation des relations entre les deux pays, et à oeuvrer pour une solution politique dans la région qui puisse permettre à la paix de s'installer durablement Il est vrai que l'Azerbaïdjan a rompu le cessez-le-feu conclu le 9 novembre 2020 avec l'Arménie à deux reprises- une première fois au début du mois d'août et, plus récemment, dans la nuit du 12 au 13 septembre l'Azerbaïdjan a fait le choix de l'emploi de la force plutôt que de la voie diplomatique pour négocier avec l'Arménie les conditions d'une paix durable au Haut-Karabagh. Il est faux de dire que la France demeure inactive, puisque, à la suite de cette nouvelle offensive, elle a demandé au Conseil de sécurité de l'ONU, qu'elle présidait alors, de se réunir. Avec le soutien de la Turquie, l'Azerbaïdjan a contraint l'Arménie à abandonner la route existante par le couloir de Latchin- étroite bande de cinq kilomètres qui relie le Haut-Karabagh à l'Arménie. Le Haut Représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a appelé à la retenue. Il faut veiller à ne pas mettre en échec les négociations engagées à Bruxelles entre les deux parties, sous l'égide de l'Union européenne, depuis quelques mois. S'il est vrai que nous importons beaucoup de gaz d'Azerbaïdjan depuis le début de la guerre en Ukraine, cet intérêt économique ne doit pas être retenu comme le déterminant majeur de l'action de la France, pays des droits de l'homme, qui a toujours su prendre et tenir des engagements courageux. Une résolution réglera-t-elle plus efficacement le conflit que la diplomatie entre nos représentants ? La question est ouverte. Le groupe RDPI n'a pas cosigné cette Avec mes collègues, nous sommes hautement préoccupés par la situation dans le Haut-Karabagh et nous condamnons fermement les graves incidents survenus dernièrement dans le secteur du couloir de Latchin.

ôterait à la France la possibilité de jouer un rôle de médiation en vue de l'établissement d'une paix durable. Bien entendu, notre groupe appelle au cessez-le-feu, au repli des forces azéries et au respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie. Au vu de ces éléments factuels, mais aussi stratégiques, la majorité du groupe RDPI a décidé d'opter pour une abstention constructive. Elle ne nie pas l'urgence, mais elle émet de sérieux et profonds doutes sur l'opportunité d'une telle proposition de résolution.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la diplomatie parlementaire est précieuse. Elle permet à des élus de discuter en toute bienveillance et de partager leurs espoirs, leurs doutes et leurs angoisses. Le groupe d'amitié France-Arménie du Sénat, que j'ai l'honneur de présider, et qui est l'un des plus actifs de la Haute Assemblée, grâce à l'engagement de tous ses membres, entretient avec son homologue de l'Assemblée nationale arménienne des relations suivies et empreintes d'une profonde et réciproque fraternité. Nos amis députés arméniens nous ont livré avec une grande franchise leurs réflexions sur la situation de leurs pays, par le passé- et notamment en 2019 -, ils nous ont alertés sur les risques d'une agression militaire. Leurs craintes étaient fondées, nous les avons relayées auprès des autorités françaises, mais elles n'ont pas été entendues. Lors de notre dernière rencontre à Erevan, en septembre dernier- je remercie ici Brigitte Devésa, Étienne Blanc et Pierre Ouzoulias de leur présence et de leur engagement tous les quatre, été bouleversés par leur désespoir et leur désespérance. Abandonnée par la Russie, oubliée par l'Union européenne et meurtrie par le voyage de la présidente de la Commission européenne à Bakou, l'Arménie leur semblait perdue.

de résolution qui nous réunit aujourd'hui n'est pas un pamphlet contre l'Azerbaïdjan ou un éloge de l'Arménie. Il s'agit de défendre la paix et nos valeurs démocratiques. Nous participons à des groupes d'amitié, non pas pour le plaisir de découvrir de nouveaux pays ou de les visiter, mais pour oeuvrer au renforcement des liens qui nous unissent et attester des difficultés C'est donc avec une certaine solennité et le devoir moral de témoigner du sentiment d'urgence absolue qui occupe les esprits de nos collègues parlementaires que je m'adresse aux trente-neuf membres du groupe d'amitié France-Arménie, à l'ensemble de notre assemblée et, bien sûr, au gouvernement français. L'Arménie a besoin de nous, de notre attention et de notre soutien ! Mes chers collègues, sachez que même dans le plus petit village d'Arménie, notre dernière résolution a été entendue et reçue avec espoir. Dans les décombres d'une petite maison de la campagne de l'Artsakh en décembre 2020, où j'ai été accueilli avec ce qu'il restait- quelques pommes et du pain -, un homme m'a dit à propos de la résolution du Sénat : « La France pense encore à nous, nous vivons encore ! ! » Non, jamais une résolution parlementaire ne consolera la souffrance des familles des disparus ! Jamais elle ne fera oublier la désolation des cimetières où les visages de soldats- si jeunes Jamais elle ne ramènera l'allégresse dans ces vignes et ces vergers ravagés par la guerre. Jamais elle ne séchera les larmes de ces populations chassées des terres de leurs ancêtres. Jamais elle ne ramènera dans son foyer le jeune qui a donné sa vie pour que triomphe dans cette partie du monde la démocratie ! Mes chers collègues, soyons certains que dans toute l'Arménie le vote de notre Sénat est attendu comme un message d'espoir par un peuple tant de fois meurtri par les catastrophes de l'histoire et qui aspire- encore plus aujourd'hui - à vivre en paix pour poursuivre son destin sur et dans ses terres.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord je tiens à remercier les présidents Retailleau et Cambon d'avoir pris l'initiative de cette proposition de résolution, ainsi que le président Marseille, qui apporte, par sa cosignature, le soutien de notre groupe.

Le Sénat a toujours été au rendez-vous lorsqu'il s'est agi de défendre l'Arménie et les Arméniens- je pense notamment à notre vote à la quasi-unanimité de la proposition de résolution portant sur la nécessité de reconnaître la République du Haut-Karabagh en 2020. Deux ans après la signature du cessez-le-feu conclu entre Bakou et Erevan, le conflit n'est toujours pas résolu et la situation reste extrêmement tendue. Alors que les regards du monde entier demeurent rivés sur le conflit ukrainien, il est urgent d'agir dans la région du Sud-Caucase.

sans grand espoir -de contenir l'escalade. Du côté de Washington, la semaine dernière, Antony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a réuni les ministres des affaires étrangères des belligérants. Du côté européen, Charles Michel et Emmanuel Macron ont été à l'initiative d'une mission d'observation qui a conclu naturellement que l'Azerbaïdjan avait mené des attaques agressives contre l'Arménie. La particularité La particularité de ce conflit est que les puissances cherchent à se poser en médiatrices, mais en faisant primer la concurrence sur la collaboration,

Ce qui vaut pour la Russie ne vaut-il pas également pour l'Azerbaïdjan ? Les efforts de sobriété que nous nous imposons pour rendre efficientes nos sanctions ne peuvent-ils pas s'appliquer aussi au régime azéri ? En 2020, des milliers d'Arméniens ont péri lors de la guerre du Haut-Karabagh. Allons-nous laisser ce conflit s'enliser ainsi ? Nous devons prendre nos responsabilités, et vite ! La France a toujours été aux côtés des Arméniens, pris en étau entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Si nous n'agissons pas, nous serons coupables et nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, par cette proposition de résolution, le Sénat honore un engagement ancien de la France en faveur de la protection des pays et des communautés chrétiennes du monde, qui aujourd'hui font, hélas ! l'objet de persécutions. Les rapports entre la France et l'Arménie s'inscrivent dans cette longue histoire que Charles de Gaulle résumait par ces mots simples : « Il y a un pacte vingt fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. » Pourquoi donc protéger l'Arménie ? D'abord parce que c'est une démocratie dans un océan de dictatures violentes : la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran- pays frontaliers de l'Arménie -violent les droits humains fondamentaux, qui sont le socle même de notre civilisation. Épuration ethnique, génocide, instrumentalisation de la justice, violence, voilà leurs outils quotidiens d'exercice du pouvoir Mais l'Arménie, elle, n'est pas dans ce camp-là, il s'en faut. C'est la raison pour laquelle il faut protéger cette si petite démocratie dans cette région du Caucase.

au petit peuple arménien ni à son armée, qui n'a du reste pas été protégée par les lois de la guerre inscrites dans la convention de Genève. L'inhumanité du président Aliyev l'a conduit à exposer dans un parc de Bakou les trophées sanglants, les casques et les vêtements de ces jeunes Arméniens, des gamins de 20 ans massacrés par l'armée d'Azerbaïdjan- victorieuse

Enfin, il nous faut protéger l'Arménie, car elle est devenue le jouet d'une rivalité géopolitique qui se dessine dans la région entre la Russie et la Turquie,

Mais protéger l'Arménie, c'est aussi nous protéger nous-mêmes face au fondamentalisme d'un islam politique totalitaire qui nie l'altérité, élimine ce qui ne lui est pas semblable. La France doit alors être du côté de l'altérité, du respect des différences, de la protection des minorités, tout cela sous couvert de la défense de la liberté de penser, de croire ou, tout simplement, de la liberté de vivre. Oui, ce que vit aujourd'hui l'Arménie, c'est ce que nous pourrions être appelés, demain, à connaître, si nous ne défendons pas ces valeurs universelles auxquelles nous croyons. Cette proposition de résolution contient trois réponses à une question que j'ai posée au Gouvernement le 5 octobre Elle propose, d'abord, de désavouer la Commission européenne, qui, sous le nom de Mme von der Leyen, a signé un accord indigne, honteux, avec l'Azerbaïdjan pour s'assurer de livraisons de gaz et de pétrole. La France ne peut pas accepter que soit sacrifiée la liberté du peuple arménien pour préserver son confort hivernal. En cela, la proposition d'embargo sur le gaz et le pétrole est sans doute une réponse à la hauteur des crimes qui ont été commis par l'Azerbaïdjan. Cette résolution monsieur le ministre, à renforcer les capacités défensives de l'Arménie en lui fournissant les armes nécessaires à sa protection. Il est temps, sur ce sujet, de passer de la parole aux actes pour protéger ce territoire, que l'on sait si fragile.

il faut que la France profite de la présidence française du Conseil de sécurité pour mettre en place la force d'interposition tant attendue. Elle garantira la souveraineté de l'Arménie sur son territoire et ses frontières, la liberté de son peuple et l'intégrité des Arméniens du Haut-Karabakh,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la dignité d'un peuple réside avant tout dans sa souveraineté et le respect de l'intangibilité de ses frontières. Le peuple arménien en est la parfaite illustration. Ce peuple, d'un courage exemplaire, se bat seul, isolé du reste du monde, dans une forme d'indifférence, contre une coalition azérie-turque et ses mercenaires djihadistes,

est de notre responsabilité première de la secourir, de la protéger, et notre inaction dans ce domaine est purement inacceptable et suicidaire. L'histoire des hommes, c'est d'abord et avant tout l'histoire des civilisations, et celles-ci, par essence, peuvent être mortelles. Or le peuple arménien, premier État chrétien du monde, appartient plus qu'aucun autre à notre civilisation et partage nos racines judéo-chrétiennes.

le cadre de la politique étrangère de l'Europe, mais également de la part de la France. Nous avons infligé d'énormes sanctions à la Russie après son agression de l'Ukraine- il fallait bien évidemment le faire -, jusqu'à renoncer à nous alimenter en gaz russe. Mais, mes chers collègues, qu'avons-nous fait concrètement pour nos amis arméniens ? En réalité, disons-le, assumons-le : pas grand-chose ! Nous nous sommes contentés, jusqu'à présent, de simples communiqués de protestation, de badge à la boutonnière, qui, malheureusement, n'ont eu aucun effet chez les agresseurs, qui sont véritablement dans une logique non pas d'apaisement, mais d'épuration ethnique, entamée avec le génocide Pis encore, Mme von der Leyen s'est rendue en personne à Bakou pour célébrer en grande pompe un nouvel accord gazier le doublement des importations de gaz en provenance de l'Azerbaïdjan. C'est purement immoral et abject ! Y aurait-il une hiérarchie dans les conflits ?

ce vieux pays dont la voix singulière vient du fond des âges. Choisir comme fournisseur de gaz l'Azerbaïdjan pour pallier le manque d'approvisionnement russe est non seulement une preuve de renoncement à nos valeurs, mais aussi, et surtout, une immense faute géopolitique, car cet accord renforce le régime autocratique, dictatorial d'Aliyev. De surcroît, cette décision européenne alimente l'ambition impérialiste de M. Erdogan, qu'il déploie depuis plusieurs années, à travers notamment une stratégie de déstabilisation internationale. Pour conclure, mes chers collègues, la question qui se pose, en fait, à travers cette proposition de résolution, est de savoir si l'Europe et la France sont prêtes à accepter, à leurs portes, un nouvel empire ottoman, plus islamique que jamais, un nouveau tyran qui, du Caucase à la Méditerranée, imposerait ses visions. En quelque sorte, est-on prêt à accepter pour quelques mégawattheures la disparition d'un peuple qui nous supplie à genoux de l'aider ? Qui oserait répondre par l'affirmative à cette interrogation ? Nous vous proposons, par cette proposition de résolution, d'envoyer un message clair et fort, de répondre non à cette question, avec la plus grande fermeté, et de défendre l'identité et la souveraineté d'un État. Il y va de notre civilisation, de notre culture et de nos racines.

d'excuser l'absence de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui accompagne actuellement le Président de la République au G20 en Indonésie. C'est donc le ministre délégué auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères qui portera la parole du Gouvernement. La proposition de résolution qui est débattue aujourd'hui devant votre assemblée porte sur un enjeu particulièrement important pour la France, pour l'Europe, et prend une acuité particulière après l'agression russe en Ukraine, au mépris de tous les principes du droit international. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, l'Ukraine subit une vague de bombardements massifs, visiblement sans précédent par son intensité, et touchant les infrastructures énergétiques de plusieurs villes d'Ukraine. La guerre, qui est revenue en Europe par l'agression russe, n'est pas sans conséquence dans la région du Caucase, qu'elle contribue à déstabiliser. Elle n'est pas sans conséquence pour l'Arménie, qui en subit le contrecoup face au défaut de légitimité d'une Russie guerrière pour se poser en faiseur de paix. Ce contexte porteur de risques d'embrasement nous conduit à redoubler d'efforts pour oeuvrer à des solutions permettant une paix et une stabilité durables dans le Caucase. La première condition de cette stabilité, et pour que les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan puissent progresser, est le strict respect du cessez-le-feu et le renoncement au recours à la force pour régler les différends. Lors des très graves affrontements qui sont survenus à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan les 13 et 14 septembre, la France s'est immédiatement mobilisée. Le Président de la République a été en contact avec le premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et avec le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, et a appelé à l'arrêt des combats, au respect de l'intégrité territoriale de l'Arménie et à un retrait des positions occupées par l'Azerbaïdjan. Nous avons aussi réuni le Conseil de sécurité sous présidence française à deux reprises, les 15 et 16 septembre, pour marquer la même exigence. Nous avons aussi obtenu l'envoi d'une mission d'évaluation de l'OSCE du côté arménien de la frontière. Aujourd'hui, c'est l'intégrité territoriale de l'Arménie qui est en jeu et qui doit être défendue. Il n'y aura pas de solution durable sans respect des principes du droit international. Aussi, l'un des objectifs majeurs du Président de la République, lorsqu'il a réuni à Prague, aux côtés de Charles Michel, le premier ministre Pachinian et le président Aliyev, a été que les deux pays confirment leur attachement à la Charte des Nations unies et à la déclaration d'Alma-Ata de 1991, par laquelle ils reconnaissaient mutuellement leur intégrité territoriale et leur souveraineté. L'autre résultat majeur de la réunion de Prague a été la mise en place d'une mission civile de l'Union européenne le long de la frontière, avec laquelle l'Azerbaïdjan a accepté de coopérer. Cette mission s'est déployée dès le lendemain du sommet de Prague pour une durée de deux mois. L'objectif de cette mission est d'établir la confiance et, par ses rapports, de contribuer aux commissions de délimitation des frontières. Son déploiement a déjà contribué à une diminution significative des incidents et des tensions. Saluons l'extrême célérité avec laquelle l'Union européenne a été en mesure de déployer ses observateurs. Et c'est à Prague, enfin, qu'a eu lieu la rencontre historique entre le premier ministre Pachinian et le président turc Recep Erdogan, grâce à l'intermédiation du Président de la République, Emmanuel Macron. La France n'a pas non plus ménagé ses efforts en faveur de la libération des prisonniers de guerre arméniens. Grâce aux interventions conjuguées de la France, de l'Union européenne et des États-Unis, trois libérations successives de prisonniers sont intervenues cette année. Nous continuons d'appeler à ce que tous les prisonniers- je dis bien tous ! -soient remis en liberté. La France est donc pleinement mobilisée dans ses efforts de médiation aux côtés de l'Union européenne, mais aussi des États-Unis, afin de parvenir à des solutions négociées sur l'ensemble des questions en suspens. Lors d'une réunion le 7 novembre à Washington, une première session de négociations s'est tenue entre les parties sur un projet de traité de paix. Nous les encourageons à poursuivre ces négociations de bonne foi,

et d'essayer de contribuer à un climat de confiance, et non de prendre des mesures de rétorsion à l'égard d'une partie, au risque de renforcer les hostilités. Il existe aujourd'hui une opportunité pour parvenir à la paix, qui doit être saisie. Ce que nous demande aujourd'hui l'Arménie, c'est de continuer à être un médiateur actif sur tous ces sujets. C'est le message que le ministre arménien des affaires étrangères m'a donné la semaine dernière- dans mon bureau -et qui guide notre action. La France continuera également d'oeuvrer au règlement de la question du Haut-Karabakh, qui demeure en suspens. Là encore, je vous invite à bien écouter ce que dit le gouvernement arménien et ce que m'a répété le ministre Ararat Mirzoyan Ararat Mirzoyan : « La question du Haut-Karabakh n'est pas une question de territoire, mais de droit. Si, dans le passé, nous placions la question du statut au fondement, en faisant dériver de lui les garanties de sécurité et les droits, désormais, nous plaçons les garanties de sécurité et les droits à la base, en en faisant découler le statut. » Ces propos courageux, le premier ministre Pachinian devant le Parlement arménien le 13 avril dernier, ont ouvert un espace de négociations, visant à définir le contenu de ces droits et de ces garanties. La France soutient cette approche, car il ne lui appartient pas de prétendre mieux savoir que le gouvernement arménien ce qui est dans l'intérêt de l'Arménie.

C'est ainsi que nous serons utiles et solidaires de l'Arménie. Mesdames, messieurs les sénateurs, aucun pays, sur la scène internationale, ne fait davantage que la France pour soutenir l'Arménie.

C'est notre devoir, notre honneur, notre fierté. C'est aussi notre combat pour la paix. Je puis vous assurer que nous poursuivrons nos efforts de médiation jusqu'à l'instauration d'une paix durable. La discussion

Je vous remercie,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, « je souhaite accompagner, encourager les initiatives, supprimer les verrous encore trop nombreux qui contraignent les territoires dans leur souhait de s'organiser mieux, en vue d'une action publique plus efficace. « Cette liberté sera laissée aux élus locaux, en lien avec les représentants de l'État aussi, pour expérimenter de nouvelles politiques publiques, de nouvelles organisations des services publics, mais aussi pour innover en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et pour définir notre territoire de demain. » Ces propos, madame la ministre, je les emprunte au Président de la République. Ils datent d'il y a cinq ans. ans. Ils ont été prononcés ici même, au Sénat, lors du lancement de la Conférence nationale des territoires. La suite, malheureusement, nous la connaissons

Les premières déclarations du Président de la République, réaffirmant une volonté décentralisatrice, les mots que Mme la Première ministre a à cette tribune, nous rappelant qu'il était nécessaire d'engager un combat pour les territoires afin de mieux entendre la voix des départements, des régions et de l'ensemble des élus locaux, sont malheureusement, après quelques semaines, restés lettre morte.

au filet de sécurité, dans lequel beaucoup de maires se sont déjà pris les pieds, considérant qu'il n'apportera qu'une aide très partielle et sommaire, voire qu'il contient des dispositifs bien trop complexes et pas du tout à la hauteur des enjeux financiers. Je pense encore aux amortisseurs sur l'énergie,

nos collectivités sont confrontées. Je le dis avec gravité et solennité : ce débat, que je remercie le groupe Les Républicains d'avoir inscrit à l'ordre du jour du Sénat,

je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour prendre part à ce débat sur la situation et les perspectives des collectivités territoriales dans notre pays, débat organisé à la demande du groupe Les Républicains.

Face à cette situation, notre gouvernement a agi sans tarder, pour les aider dans l'urgence, mais aussi pour qu'elles maintiennent leurs capacités d'investissement, en particulier en faveur de la transition écologique. écologique. Nous n'avons pas construit ces mesures dans un exercice solitaire. Conformément à notre engagement, nous n'avons cessé d'échanger avec les associations d'élus, pour tenir compte de leurs remontées de terrain et de leurs propositions.

volet est l'aide concrète apportée aux collectivités face à l'inflation. Grâce au filet de sécurité, 1,5 milliard d'euros sont mobilisés pour l'ensemble des collectivités fragilisées par l'augmentation des dépenses d'énergies. ajouter à ce montant les moyens dédiés au bouclier tarifaire, ainsi qu'à « l'amortisseur électricité », soit plus de 1 milliard d'euros, qui conduiront à alléger les charges liées à la hausse de l'électricité pour toutes les collectivités.

la dotation de solidarité rurale (DSR). Cela permet à 95 % des communes de voir leurs dotations maintenues ou augmentées. Ce renforcement de la DGF est couplé à la pérennisation de l'ensemble des dotations d'investissement- dotation de soutien à

Ces dispositifs ont été amendés, modifiés et perfectionnés à l'Assemblée nationale pour être adaptés aux besoins des collectivités. Vous aurez l'occasion de les améliorer encore dans le cadre de votre examen du texte, j'imagine. Notre volonté de dialogue est sincère. les perspectives des collectivités territoriales se trouvent également les programmes d'appui que nous mettons en oeuvre depuis le précédent quinquennat. Nous poursuivrons

Je viens de finaliser l'acte II d'Action coeur de ville, pour accentuer encore son élan, avec la volonté de soutenir davantage des projets de valorisation liés à la transition écologique.

Notre objectif est aussi d'élargir encore le cercle de nos partenaires. Plus largement, nous poursuivrons dans la dynamique de l'agenda rural, au sein duquel s'inscrivent ces deux mesures. permis d'améliorer concrètement la qualité de vie de nos concitoyens dans les communes rurales, en particulier en matière de proximité des services publics, avec les espaces France Services. Il en existe déjà plus de 2 400 dans tout le pays ; il y en aura 2 600 à la fin de l'année.

Cette liste de programmes d'appui n'est pas exhaustive, mais il me semble important de souligner la continuité de notre action, ainsi que notre exigence de méthode. Dans l'ensemble de ces dispositifs, l'État se fait en effet accompagnateur et non prescripteur, au service des projets portés par les élus locaux, notre but est une plus grande efficacité au bénéfice de tous. Nous les améliorons à la lumière des retours d'expérience, et vous êtes d'ailleurs nombreux à contribuer à cette démarche.

Nous mettons également en place le remboursement forfaitisé des frais de garde des élus, une mesure qui facilitera grandement la vie quotidienne des intéressés. Il leur suffira de déposer un dossier de remboursement des frais réels.

d'une avancée supplémentaire pour garantir aux élus locaux un exercice serein de leur mandat. Mesdames, messieurs les sénateurs, vous le voyez, le Gouvernement s'engage résolument aux côtés des élus locaux et des collectivités.

Le Gouvernement dispose pour répondre d'une durée équivalente. Il aura la faculté, s'il le juge nécessaire, de répondre à la réplique pendant une minute supplémentaire. L'auteur de la question disposera alors à son tour du droit de répondre pendant une minute.

le 49.3, vous vous permettez d'imposer de façon cavalière, sans discussion préalable, l'encadrement renforcé des dépenses de fonctionnement pour un certain nombre de collectivités territoriales. Cet encadrement des

ces nouveaux contrats ou, au contraire, instaurer un véritable dialogue pour construire les réponses indispensables pour aujourd'hui comme pour demain et, ainsi, développer les territoires de notre République

la dette française. Il est donc nécessaire que le Gouvernement et le Parlement montrent clairement qu'ils font cet effort. C'est le sens des trajectoires budgétaires qui sont inscrites en loi de programmation des finances publiques. Le pacte de confiance est-il le meilleur outil Il est, à mon sens, bien plus responsabilisant pour les collectivités que les mécanismes précédents. Je rappelle, à ce titre, que sous le mandat de François Hollande l'État avait autoritairement baissé la DGF de plus de 11 milliards d'euros en guise de trajectoire. Pour autant, ce pacte peut évidemment être amélioré, et le rôle des collectivités dans cet effort pourrait se manifester autrement. Je suis ouverte au dialogue et je compte sur la sagesse du Sénat pour formuler des propositions.

Chacun sait ici de quoi il est question : certains d'entre nous parce qu'ils étaient déjà sénateurs en 2010, lors de l'examen de la loi de réforme des collectivités territoriales, dite RCT, acte de naissance du conseiller territorial, d'autres- c'est mon cas -, parce qu'ils étaient alors élus locaux, donc concernés par cette réforme.

La région Normandie, qui m'est particulièrement chère, ne compte pas moins de 262 élus départementaux. Avec le conseiller territorial version 2023, ces 262 élus constitueraient-ils le nouvel effectif du conseil régional, qui n'a aujourd'hui que 102 membres ?

À quelle échéance envisagez-vous une telle réforme ? Enfin, la Première ministre évoque l'idée de « simplifier le millefeuille territorial ». conseiller territorial annonce-t-il la disparition à terme d'un niveau de collectivité, comme certains le craignaient en 2010 ? La parole est à Mme

Rassurez-vous : si votre crainte porte sur l'avenir des conseillers départementaux, le conseiller territorial ne marquera pas la fin des départements. est au contraire de permettre au territoire de recevoir de meilleurs services publics de la part des collectivités départementales et régionales et aux élus d'être

est à M. Stéphane Ravier. Madame la ministre, pour les collectivités territoriales, la crise n'est pas une surprise. Elles subissent les erreurs des gouvernements dans la politique énergétique, leur soumission aux diktats de l'Union européenne et leur incapacité à miser sur une décentralisation effective. Arrêt programmé des centrales nucléaires, obligation pour EDF de racheter plus cher l'électricité qu'elle a vendue, sanctions contre la Russie mettant en difficulté les ménages français : à la roulette de l'idéologie, c'est le Gouvernement qui joue et les collectivités qui perdent et qui paient. Les maires ne font plus de choix ; ils sont contraints en tout et cherchent des solutions de sauve-qui-peut.

Le choix est fait d'éteindre l'éclairage public au coeur de la nuit dans de nombreuses communes ; c'est un blackout communal contraint, avant qu'il ne soit subi et soudain. À Sénas, les crèches, la gestion des espaces vert et les cantines sont en régie municipale, et l'on réfléchit à ne pas conserver la totalité du personnel. Les autres échelons de collectivités étant aussi touchés, les communes ne peuvent plus compter sur leur concours. Par exemple, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il n'y a plus assez d'aides de la région pour financer des équipements et des constructions, car la facture du chauffage des lycées est passée de 17 millions d'euros Les solutions se trouveront dans une décentralisation de la fiscalité et dans un retour du consentement à l'impôt par la démocratie de proximité. Cette crise est un révélateur de la traversée du désert des collectivités depuis des années, comme la crise du covid-19 a mis à nu un hôpital rongé par l'austérité unilatérale. Je n'ai rien entendu dans vos propos, madame la ministre, qui annoncerait une prise de conscience de l'État : rien sur le retour à une souveraineté nationale qui protège, rien sur une baisse des coûteuses et inutiles dépenses publiques de l'État. quelle est votre stratégie à moyen terme pour permettre l'autonomie fiscale des collectivités et pour sauver les services de proximité par une véritable décentralisation ?

à la demande des associations d'élus, ou encore le renforcement de la dotation de biodiversité. Toutes les collectivités seront éligibles à l'amortisseur électricité annoncé par la Première ministre, et 1 milliard d'euros seront pris en charge par l'État à ce titre. Les collectivités les plus fragiles pourront bénéficier du filet de sécurité sur leurs dépenses d'énergie, une aide de 1,5 milliard d'euros assumée par l'État, en plus des 430 millions d'euros de 2022. Enfin, les marges préservées devront permettre aux collectivités d'investir. Là aussi, l'État est présent à leurs côtés 2 milliards d'euros pour les investissements, qui est doublée grâce aux 2 milliards d'euros du fonds vert. Quant au nouvel acte de décentralisation, le Président de la République a fixé son cap le 10 octobre dernier. Sa volonté est claire : allier compétences, moyens et responsabilités. Le format et le calendrier des réflexions et de la nécessaire concertation seront précisés. Un cadre existe déjà pour échanger sur les sujets structurants de notre action commune, à par la commission transpartisane sur les institutions, annoncée par le Président

L'inverse est-il vrai ? Là où se trouvent de grandes responsabilités, trouve-t-on de grands pouvoirs ? L'adaptation au changement climatique et la sécurisation des populations face à ces risques répétés et mortifères constituent l'un des plus grands défis auxquels nos collectivités devront faire face Dans ce contexte, les communautés de communes rurales et de montagne qui disposent de nombreux linéaires d'eau susceptibles de déborder ont, depuis le 1 janvier 2018, la grande responsabilité de la prévention des inondations en exerçant la compétence de (EPCI) sont, comme toutes les collectivités locales, touchés de plein fouet par l'inflation. Ils prennent en charge l'augmentation du point d'indice de nos fonctionnaires et font face à des factures énergétiques salées.

Madame la ministre, l'entretien nécessaire des ouvrages et la sécurisation des personnes et des biens passent aujourd'hui au second plan, faute de capacités d'investissement de ces EPCI. Pis encore, le risque est aujourd'hui certainement minoré. Rappelons que l'article 56 de la loi Maptam prévoit le transfert dès 2024 de l'entretien des ouvrages de prévention des inondations aux autorités « gemapiennes

horizontale. La loi 3DS, a ouvert le champ de la différenciation territoriale. Il est temps d'y ajouter celui de la solidarité. Madame la ministre, quand allez-vous proposer une réforme du financement du risque d'inondation lié aux cours d'eau prévoyant un véritable partage de la responsabilité ? Comptez-vous repousser le transfert de responsabilité prévu pour

les EPCI à fiscalité propre exercent la compétence Gemapi et doivent, à ce titre, gérer les ouvrages de protection contre les inondations. Dans une période transitoire, qui doit donner aux acteurs le temps de s'organiser, l'État gère certains ouvrages jusqu'en 2024. Le transfert représentera indéniablement un investissement important pour les collectivités, mais plusieurs outils financiers sont déployés pour accompagner ces dernières. le fonds de prévention des risques naturels majeurs appuie jusqu'en 2027 les études et les travaux sur les anciennes digues de l'État. La taxe Gemapi permet en outre de prélever jusqu'à 40 euros Ensuite, 2 milliards d'euros sont disponibles au titre des financements des agences de l'eau et du dispositif Aqua Prêt, géré par la Caisse des dépôts. Enfin, la loi 3DS rend possible une expérimentation destinée à mieux associer les établissements publics territoriaux de bassin à cette politique par des financements dédiés ; elle permet en outre aux EPCI de se regrouper dans des structures dédiées, afin d'atteindre la bonne échelle de gestion hydrographique.

de nos territoires, particulièrement de nos communes, et, en l'espèce, de celles de mon département. En effet, elles sont nombreuses à avoir récemment délibéré sur les conséquences de la crise financière et économique, qui fragilise leur budget, et je partage bien évidemment leurs inquiétudes.

Décentraliser la gouvernance de cette dotation conduirait donc à diluer la cohérence et l'efficacité des politiques publiques sous-jacentes.

au fonds vert, il bénéficiera d'une gestion souple, proche des territoires, sans appel à projets ni à manifestation d'intérêt. Les crédits seront délégués au préfet du département, les enveloppes seront fongibles et les financements orientés vers des projets locaux soutenus soutenus par les élus. Le Fonds pourra financer un certain nombre de politiques publiques, notamment la rénovation énergétique des bâtiments ou encore le renouvellement de l'éclairage public.

partout en France, depuis le début de la crise, les élus rivalisent d'ingéniosité pour trouver de nouvelles solutions leur permettant d'éviter d'augmenter les impôts tout en maintenant les investissements. Certains ont d'ores et déjà réduit l'éclairage public et les plages horaires d'ouverture des bâtiments communaux, immobilisé une partie de leur parc de véhicules destiné aux agents

problème de la collectivité que vous avez mentionnée, dont le tarif s'élevait à 400 euros. Ensuite, pour les collectivités fragilisées par cette hausse, le filet de sécurité sera reconduit en 2023. Concrètement, si l'épargne brute de la collectivité se dégrade et si la hausse attendue des recettes fiscales ne permet pas d'absorber la hausse des dépenses d'énergies, l'État versera une compensation à la collectivité. Le coût combiné de l'amortisseur et du filet est estimé à 2,5 milliards d'euros.

le principe « qui commande paie » n'est malheureusement pas satisfaite à ce jour, pour tout un tas de raisons. La redondance des couches administratives, la politisation des moyens financiers alloués, l'inadéquation constante des dotations de l'État et la baisse des ressources fiscales locales limitent tous les jours la capacité de bonne gestion de nos communes.

vous m'interrogez sur la pérennité du financement des compétences nouvellement exercées par les collectivités et sur le modèle des finances locales, en lien avec le récent rapport de la Cour des comptes, transmis au Sénat. Vous le savez, le transfert de compétences de l'État vers les collectivités territoriales

ce choix qui a été réalisé lors de la suppression d'impôts locaux : la suppression de la taxe d'habitation communale a été accompagnée du transfert du même montant de taxe foncière ; la suppression de la CVAE s'accompagnera d'un transfert de TVA dynamique. Vous le voyez,

consiste à pousser le curseur du financement par les subventions au maximum ; un autre consiste à faire l'inverse. Je reste donc évidemment à l'écoute des propositions du Sénat, qui seront sans aucun doute nourries de ce rapport.

Durant la crise sanitaire, ces derniers ont su, chacun à son échelon de compétence, faire la démonstration de leur détermination à garantir la santé et la sécurité de leurs concitoyens.

L'enchevêtrement des compétences nuit en effet à la bonne compréhension par les citoyens de l'action publique, les en éloigne et

Elle n'excluait pas, pour y parvenir, d'instaurer un conseiller territorial. En Alsace, la mise en oeuvre d'un tel conseiller aurait tout son sens. Véritable laboratoire de l'innovation territoriale depuis les premières lois de décentralisation, l'Alsace fait aussi figure de précurseur de la différenciation chère au Président de la République, puisqu'elle a créé la Collectivité européenne d'Alsace. Le Gouvernement serait-il prêt à engager une réflexion sur la mise en oeuvre de ce conseiller territorial dans le territoire alsacien ? À titre expérimental, avant son éventuelle extension au reste du territoire, ce conseiller exercerait, dans le périmètre alsacien, les compétences de la Collectivité

pour notre organisation institutionnelle. Le calendrier et le format de cette concertation annoncée par la Première ministre seront précisés très prochainement. L'Alsace et le Grand Est seront, au même titre que l'ensemble des départements et régions,

C'est aussi une condition de la démocratisation des fonctions électives, dans un contexte de technicisation du gouvernement local. La formation des élus locaux a connu des réformes : certaines utiles, d'autres guidées par la maîtrise des coûts.

Le 25 octobre dernier, l'exercice s'est encore durci, avec la mise en place d'une authentification numérique renforcée, FranceConnect+, pour accéder à Mon compte élu.

Alors qu'un préavis avait été demandé, ce basculement a finalement eu lieu sans information préalable des élus locaux et sans délai, symptôme supplémentaire de la défiance existant entre l'État et les collectivités.

Le non-recours pourrait ainsi devenir la règle et priver les élus du bénéfice de la formation. Après deux années de « surmobilisation » du Dife, le système de formation connaît une crise, en dépit de l'enjeu important de massification de la formation. Le rapport de gestion de la Cour des comptes dénombre 32 000 formations financées en 2021, contre 4 029 de janvier à fin août 2022 ... Madame la ministre, qu'entendez-vous faire pour faciliter la formation des élus locaux ? Quelles améliorations envisagez-vous d'apporter à Mon compte élu, pour que ce service soit un service adapté et que les organismes de formation puissent accompagner

ont d'ores et déjà permis de rétablir financièrement le système et d'aboutir à une modernisation des pratiques. La plateforme Mon compte élu permet de mieux informer les élus, qui disposent dorénavant de l'ensemble

enceinte, n'a pas été contacté par SMS ou par téléphone sur ce sujet ? Mes services ont fait en sorte que l'accès à la formation des élus locaux ne soit pas restreint

dans les maisons France Services ou à domicile. Nos contacts avec les associations d'élus et le secteur de la formation sont réguliers, afin d'entendre les difficultés qui pourraient se faire jour et d'améliorer les choses là où c'est nécessaire.

» Madame la ministre, sans préjuger des résultats de la concertation que vous avez annoncée et du travail conduit par le Sénat sous l'autorité du président Larcher, pouvez-vous nous exposer votre vision et celle du Gouvernement

de répondre imparfaitement aux attentes de nos concitoyens. Ce travail doit être une oeuvre collective. Tel est le sens de la commission transpartisane qui sera prochainement instituée. J'imagine que les sénateurs y prendront toute leur part. C'est également la dynamique enclenchée par le Conseil national de la refondation et ses déclinaisons territoriales et thématiques.

potentiellement structurants pour notre organisation territoriale. La concertation est le fil conducteur de notre action, et ce partenariat avec les élus est incontournable, essentiel.

donnons tout son sens à la loi 3DS, avec une application territorialisée, qui permettra d'avancer au plus près des attentes des des différents territoires, parce qu'il ne se passe pas la même chose dans les Bouches-du-Rhône et dans le Nord ou le Pas-de-Calais. Si l'on utilise bien la loi 3DS, on pourra enregistrer des avancées, dans l'intérêt des territoires.

part, le contexte économique se dégrade, avec notamment la hausse du prix de l'énergie et des matières premières, l'augmentation des taux d'intérêt fait peser une lourde menace sur une recette stratégique pour nombre de départements : les ailleurs, il est établi que le marché de l'immobilier est cyclique et que les départements sont exposés aux évolutions de l'économie de façon procyclique. Ainsi voit-on se profiler le redoutable effet de ciseaux bien connu, alors que les départements sont privés de tout levier fiscal pour affronter des difficultés que l'on espère conjoncturelles, comme ils ont pu le faire à la suite de la crise financière de 2008-2009.

donc vous demander, madame la ministre, comment vous comptez sécuriser plutôt que fragiliser les finances départementales. Êtes-vous favorable à une loi de finances entièrement consacrée aux finances locales ? La parole est à Mme la ministre

leur facture d'électricité et le filet de sécurité sera étendu aux départements et aux régions, contrairement à ce qui s'est

de vente de l'électricité au bénéfice de toutes les collectivités, quelle que soit leur taille ; troisièmement, et enfin, le relèvement du plafond de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, qui amortit la volatilité du marché.

de recettes, les communes ultramarines profiteront également de la hausse de la DGF en 2023, laquelle sera renforcée par rapport à l'Hexagone du fait de l'augmentation de la

à la progression automatique des dotations. Tel est le complément d'information que je voulais vous apporter, madame la sénatrice.

à 5,5 %, atteint son niveau le plus haut depuis 1985. L'augmentation du point d'indice de 3,5 %, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, représente 2,3 milliards d'euros. La baisse des dotations se poursuit avec le gel de la DGF depuis 2017. depuis 2014, la baisse cumulée des dotations aux collectivités représente 46 milliards d'euros, ce qui a conduit à l'effondrement des investissements. À cela s'ajoutent, dans le projet de loi de finances pour 2023, la suppression de la CVAE et le fameux pacte de confiance, lequel encadre les dépenses d'un grand nombre de communes.

Avec une croissance annoncée à 1 % en 2023, l'urgence est de soutenir l'investissement public local, en particulier en accompagnant la transition écologique des transports et des logements.

de maintenir l'indexation des bases fiscales, de revoir les modalités de la suppression de la CVAE, de renoncer à tout dispositif d'encadrement de l'action locale de sorte à éviter une perte de 15 milliards d'euros,

Madame la ministre, quelles mesures proposez-vous pour redonner de la lisibilité, de l'efficacité et de la confiance aux maires et aux présidents d'intercommunalités, assurant ainsi l'autonomie fiscale et la libre administration des collectivités locales et territoriales ?

et les départements. Cette compensation a fait l'objet d'échanges très constructifs avec les nombreux présidents d'associations d'élus. De fait, nous avons abouti à une solution qui leur convenait, c'est-à-dire une part

De plus, l'inflation alimentaire se répercute fortement sur la restauration collective ; pour la seule restauration scolaire, le surcoût est estimé à 648 millions d'euros. Dans de telles conditions, la suppression de services et d'emplois s'impose dans un nombre croissant de collectivités comme la seule solution pour boucler leur prochain budget. Aussi, l'État devrait déployer des mesures pour protéger les collectivités, comme il a su le faire pour préserver les entreprises face au covid-19. Pourtant, de manière incompréhensible, vous aggravez une telle situation, madame la ministre, par la poursuite du désarmement fiscal des collectivités au travers de la suppression de la CVAE. Après la taxe d'habitation, vous supprimeriez ainsi l'une des dernières recettes dynamiques des collectivités. Non seulement vous affaibliriez encore l'autonomie financière de ces dernières, mais vous décideriez de priver le pays d'une recette de 8 milliards d'euros, au moment même où vous appelez chacun à un effort de maîtrise des finances publiques. Vous vous étiez félicitée, notamment dans cet hémicycle, d'une méthode renouvelée dans l'élaboration du volet territorial du PLF, passant par une démarche de coconstruction avec les associations d'élus. Une telle démarche est louable. Pourtant, il semble que le budget qui en ressort ne tient pas compte des principales attentes exprimées par les élus locaux. Au-delà des moyens nécessaires pour fonctionner, les collectivités ont besoin d'une vraie relation de confiance avec l'État et d'une autonomie financière préservée. Plusieurs mesures de ce PLF tournent clairement le dos à cette attente légitime.

ménagères. Les ordures ménagères pèsent pour près de 20 milliards d'euros dans le budget de nos collectivités locales. Ces budgets annexes sont actuellement victimes de l'explosion des coûts de l'énergie et de l'inflation. En conséquence, les taxes et redevances d'enlèvement des ordures ménagères payées par les usagers augmentent fortement, ce qui pèse sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. À ces augmentations conjoncturelles s'ajoute l'aggravation de la taxe générale sur les activités polluantes Cette taxe s'alourdit au fil des années, selon une trajectoire pensée pour inciter collectivités et usagers à moins enfouir et moins incinérer. On peut comprendre et partager madame la ministre, votre collègue Mme Couillard reconnaissait devant la commission du développement durable du Sénat, la semaine dernière, que la nouvelle filière de déchets du bâtiment ne serait en place que d'ici à un an ou deux seulement, admettant, par là même, le retard pris dans la mise en place de ces filières à responsabilité élargie des producteurs. Dans l'attente, les déchets demeurent et sont ainsi soumis à la TGAP. Au regard de ces retards qui ne sont imputables ni aux collectivités ni aux usagers, il paraît plus cohérent et plus juste de décaler d'un an la prochaine aggravation de la TGAP, prévue pour 2023, le temps que des solutions de substitution soient mises en place.

des collectivités territoriales qui gèrent les déchets. De fait, le but de cette hausse de la TGAP était en quelque sorte de presser l'épée dans les reins des collectivités pour améliorer les projets de traitement de déchets et éviter, vous l'avez dit vous-même, la mise en décharge ou l'incinération. fait pas exception, nous agissons en concertation, en essayant de donner à nos interlocuteurs le plus de visibilité possible. La trajectoire d'augmentation progressive jusqu'en 2025 avait été annoncée dès 2018, si je ne me trompe, pour permettre aux acteurs de s'organiser. En outre, l'État soutient financièrement les projets de valorisation des déchets des collectivités, pour un montant de 80 millions d'euros en 2021. La baisse de la TVA sur la valorisation des déchets, elle aussi, permet aux

pour la collecte des biodéchets. Cela dit, je comprends vos interrogations. Je sais d'ailleurs que Bérangère Couillard est en contact avec les associations qui représentent les collectivités pour trouver des solutions consensuelles. En échangeant avec les collectivités et ma collègue, je m'assurerai que ce dialogue soit constructif et fructueux. Ainsi, nous verrons si nous pouvons ouvrir le débat sur un gel momentané de cette augmentation de la TGAP.

une perte de légitimité de l'action publique en découle. Ce ne devrait pas être la moindre de nos préoccupations. Alors que l'on parle de couple maire-préfet, voire de couple président d'intercommunalité-préfet, j'aimerais entendre parler de couple maire-habitant. Dans une démocratie, ceux qui décident sont ceux qui ont été choisis par le peuple ; mais les élus ne décideront bientôt de plus rien. Madame la ministre, êtes-vous prête à redonner un pouvoir d'agir plus important

les collectivités doivent faire face à des charges de plus en plus élevées, bien souvent dues à des facteurs externes sur lesquelles elles n'ont aucune maîtrise. Ces derniers mois, par exemple, la revalorisation par l'État du point d'indice de la fonction publique, la hausse de l'inflation ou l'explosion du coût de l'énergie ont fait flamber les dépenses des communes. Face à ces nouvelles contraintes budgétaires, peu de collectivités parviennent à dégager les montants suffisants pour mettre en oeuvre leurs programmes d'investissement. Bien souvent, les seuls projets qui peuvent être financés par les communes sont ceux éligibles à des cofinancements de l'État, au travers de subventions ou de portages financiers ; pensons à la DETR, dont l'attribution se fait à la discrétion du préfet. En conséquence, sans l'aval de l'État, il devient de plus en plus difficile pour un maire de mettre en oeuvre un projet pour sa commune. Ces mécanismes de plus en plus présents dans la vie communale conduisent à s'interroger sur le fonctionnement de nos institutions et sur le respect de l'esprit de l'article 72 de la Constitution garantissant la libre administration des collectivités. Cette mise sous tutelle déguisée est dure à vivre pour les élus locaux. Ils perdent peu à peu leur pouvoir décisionnaire dans un grand mouvement de recentralisation qui ne dit pas son nom.

des collectivités et l'indexation de la DGF. Je le répète, il n'y aura pas cette année de désindexation, pour des raisons financières évidentes et pour que le Gouvernement puisse respecter la trajectoire qu'il s'est fixée.

perdues ont été remplacées par d'autres recettes fiscales du même montant et de même nature. La boussole du Gouvernement est véritablement la préservation des marges de manoeuvre financières

demande. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelles sont les attentes des élus locaux, qui traduisent celles, majoritaires, de nos concitoyens ? C'est d'accéder à un pacte de responsabilité et de confiance, pour faire émerger le clair de l'obscur et dénouer le noeud gordien permettant de boucler leur budget. Cela passe, bien sûr, par un retour de l'autorité et par une meilleure reconnaissance du travail, mais aussi par une nouvelle approche territoriale. Cela ne peut reposer que sur une grande démarche décentralisatrice bâtie sur les principes de subsidiarité, de liberté et de responsabilité, établissant que chaque niveau décide de ce qu'il fait et de ce qu'il renvoie à celui du dessus, qu'il le fasse de manière libre, dans un cadre défini, c'est-à-dire dans un cadre contractuel assis sur l'autonomie financière. Rappelons à ce titre que le niveau de la dépense publique locale est bien inférieur en France à ce qu'il est dans les autres pays européens : 19 % contre 40 %. La situation des collectivités dans notre pays est contrastée. Fruit de l'histoire et de la géographie, des richesses et des initiatives, des gestions passées et en cours, la collectivité est toujours responsable. pour preuve les efforts continus pour répondre aux exigences de gestion, notamment à la règle d'or qui s'impose à elle. J'en veux également pour preuve les adaptations continues pour répondre aux attentes du quotidien en matière de services publics et d'infrastructures, de cadre de vie et de fierté locale, mais aussi pour préparer l'avenir de nos territoires renforcer leur attractivité, dans le respect des caractéristiques propres à chacun. Les perspectives sont souvent empreintes d'inquiétudes, de perte de sens, de découragement face à la bureaucratie, à l'éloignement, au manque d'écoute et de représentation et à l'explosion des dépenses énergétiques. sont aussi pleines d'envie, de volonté, d'un formidable engagement quotidien au service des autres, que je veux saluer. Beaucoup se sentent aujourd'hui « dépossédés ni en situation d'agir face à des contraintes administratives fortes et aveugles, ni en situation de faire, car leurs moyens sont comptés, ni en situation de véritablement décider face à une complexité croissante, à une intercommunalité à la gouvernance non encore adulte et à un État contraignant. En fait, notre décentralisation est pour l'essentiel administrative et non politique. On a confié des tâches aux élus et aux collectivités, mais on leur a rarement donné les moyens juridiques et financiers d'y répondre en autonomie et en responsabilité. Les attentes qui pourraient devenir des perspectives sont orientées dans quatre directions, que je n'aurai pas le temps de développer ici, mais que j'évoquerai brièvement. Premièrement, il convient de faire preuve de bon sens et de confier aux collectivités locales tout ce qui relève de la vie quotidienne. de préserver et de développer les biens communs, ce qui nécessite d'investir massivement dans les infrastructures, dans le respect de l'environnement. Troisièmement, il faut garantir à chacun le bien-être : cela consiste à réinvestir nos territoires par les services publics de proximité et, d'abord, ceux de la sécurité, de l'éducation et de la santé. enfin, donnons à tous les justes moyens d'agir, en réinterrogeant le mode de financement des collectivités territoriales. Les priorités sont de débureaucratiser, de réenraciner et bien sûr de simplifier, en limitant pour cela l'administration administrante.

Cela passe par une réelle capacité d'autofinancement des collectivités territoriales, laquelle est bien mise à mal aujourd'hui. Cela nécessite de faire preuve de courage, en garantissant la traçabilité de l'argent public, pour rendre la dépense efficace et redonner un espoir à chacun. La refonte de la procédure des marchés publics, dont chacun voit bien aujourd'hui combien elle est inflationniste, serait un véritable signe pour garantir l'investissement. Un horizon pourrait être ouvert par une réforme constitutionnelle donnant une liberté normative aux territoires, par extension de l'article 73 de la Constitution. Quelle belle perspective s'ouvrirait à chacun si ce texte ne s'appliquait plus aux seules collectivités d'outre-mer, mais à l'ensemble du territoire, ouvrant enfin la voie à l'indispensable différenciation Enfin, en matière de financement des collectivités territoriales, ce sont les libertés locales, la lisibilité, la justesse et la subsidiarité qui doivent primer. Pour cela, nous devons ouvrir ce chantier sans tabou, car, en dépit d'un consensus sur le diagnostic, les propositions de réformes, qui doivent garantir l'autonomie et la lisibilité pour les collectivités locales, évidentes. Mon collègue Mathieu Darnaud l'a rappelé, le Sénat a déjà beaucoup travaillé sur ces sujets, et il continue de le faire. Sur l'initiative de notre président Gérard Larcher, un groupe de travail s'active pour nourrir les projets du Président de la République en matière institutionnelle et territoriale, avec, comme pilier majeur, la commune. Soyez certains que notre groupe sera au rendez-vous des attentes pour redonner des perspectives. C'est une urgente exigence démocratique. Nous en

de se constituer partie civile pour soutenir pleinement, au pénal, un édile victime d'agression, présentée par Mme Nathalie Delattre et plusieurs de ses collègues (proposition n° 631

nous nous souvenons tous de Jean-Mathieu Michel, maire de la commune de Signes, dans le Var, élu depuis plus de trente ans. Nous avions tous été émus et affectés par cette nouvelle terrible. Ce qui débouchait sur des incivilités voilà encore quelques années donnait désormais lieu à un drame. Le Sénat, par l'intermédiaire de la commission des lois, présidée à l'époque par Philippe Bas, avait lancé une consultation nationale. Son rapport sur les menaces et les agressions auxquelles sont confrontés les maires est venu confirmer par des chiffres ce que chacun pressentait : 92 % des élus consultés et ayant répondu disaient avoir été victimes d'incivilités, d'injures, de menaces ou d'agressions physiques. Trois années plus tard, rien n'indique une amélioration de la situation, tant pour les maires, considérés pourtant comme « les élus préférés des Français » que pour les autres dépositaires de l'autorité publique ou de fonctions électives. J'ai une pensée particulière pour mes élus girondins : Philippe Bécheau, maire de Saint-Philippe-d'Aiguille, agressé le 5 août 2020 ; Cédric Gerbeau, maire de Saint-Macaire, agressé le 8 décembre 2021 Kilian Alliot, conseiller municipal de Sainte-Eulalie âgé de 25 ans, agressé le 16 décembre 2021 ; Patrick Gomez, maire de Sadirac, menacé voilà quelques semaines ; et tous les autres, trop nombreux pour que je les cite ici. Pour l'année 2021, les statistiques nationales dénombrent plus de mille agressions d'élus, allant du courriel de menace à l'attaque physique, soit une hausse de 50 % par rapport aux années précédentes, alors même que, nous le savons, peu d'élus portent plainte. Ce chiffre est donc bien en deçà de la réalité. Nous en venons même à former les élus pour prévenir les débordements lors d'échanges difficiles avec nos concitoyens. Maires et adjoints sont en effet les premières cibles de la violence, car ils interviennent, en proximité, sur des sujets souvent liés à des troubles de voisinage, à l'alcoolisation sur la voie publique, au tapage nocturne ou diurne, aux problèmes liés aux règles d'urbanisme, à la circulation routière ou encore aux violences intrafamiliales. Toutefois, au-delà de ces motifs concrets, l'augmentation des agressions est aussi l'expression d'un phénomène plus profond.

que « la capacité des institutions à trouver des solutions face à la crise actuelle, économique et sociale, est régulièrement mise en doute. » Ainsi, certains semblent désormais considérer que la soumission à une norme commune ne va plus de soi, ce qui justifie toutes sortes de comportements. Qu'il y ait une forme de désenchantement envers le politique depuis plusieurs années, nous pouvons l'entendre. Il est de notre responsabilité de tout mettre en oeuvre pour inverser cette tendance et y remédier. En revanche, nous ne pouvons plus accepter d'être conciliants à l'égard des agresseurs de ceux qui se dévouent à la vie démocratique de leur collectivité. Nous ne devons plus pardonner au nom de je ne sais quel sentiment de culpabilité ou de la responsabilité coûte que coûte. Nous devons toutes et tous faire preuve d'une intransigeance intégrale. Il s'agit de l'essence même du contrat social, tel que l'ont imaginé les Lumières, de Hobbes à Rousseau. La brutalité la plus primitive ne saurait être admise comme une réponse légitime dans une société républicaine. Malheureusement, cette banalisation de la violence, nous l'avons encore observée ces derniers jours, dans un média. Le parlementaire Louis Boyard a fait l'objet de nombreuses insultes. Si je suis loin de partager toutes ses idées, de partager toutes ses idées, je veux lui dire mon soutien dans sa démarche judiciaire. Rien ne justifie un tel acharnement. Et, ce qui est plus grave encore, ces images contribuent à renforcer l'impunité avec laquelle des concitoyens s'en prennent aux élus locaux. Alors, bien sûr, il existe déjà des mécanismes spécifiques pour répondre aux besoins concrets de la protection des élus. Le droit pénal permet de tenir compte de la qualité des victimes, selon qu'elles sont dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif. Ainsi, une simple insulte peut être qualifiée d'outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, plutôt que d'injure. De même, la commission de faits au préjudice d'un élu constitue une circonstance aggravante, dès lors que la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur de l'infraction et que les faits sont commis en raison de ses fonctions. C'est pourquoi il nous faut rappeler aux élus de bien décliner leurs fonctions électives lorsqu'ils interviennent auprès de personnes issues ou non de leur commune. Cependant, au-delà du droit strict, se pose surtout la question concrète de la réponse dans les tribunaux. C'est dans ce cadre qu'existent, selon moi, des carences. Dans de trop nombreux cas, malgré la récurrence des faits et leur gravité, nous observons que la poursuite judiciaire n'aboutit pas souvent. Une telle situation a constitué le déclencheur de la proposition de loi que nous étudions ce soir. Elle a été cosignée par 95 de mes collègues sénateurs, que je remercie ; Éric Gold, qui avait déposé un texte en la matière, l'a également cosignée. Le Gouvernement a d'ailleurs conscience de cette carence, puisque, dans une circulaire du 7 septembre 2020, vous avez, monsieur le garde des sceaux, procédé à un rappel auprès des procureurs. leur avez enjoint de toujours veiller à retenir des qualifications pénales applicables prenant en compte la qualité des victimes, lorsqu'elles sont dépositaires de l'autorité publique, chargées d'une mission de service public ou investies d'un mandat électif. D'autre part, vous avez insisté sur un point qui mène à l'objet même de ma proposition de loi, à savoir une réponse pénale systématique et rapide, apportée par les parquets.

Dans la plupart des cas, les plaintes sont soit classées sans suite ou ne font l'objet d'aucune suite pénale, même pas d'un rappel à la loi ou de mesures d'éloignement du territoire de la commune. Il y a donc urgence à proposer que les élus victimes soient mieux soutenus dans l'engagement d'une procédure pénale, afin que justice leur soit rendue. Pour cela, j'ai considéré, en travaillant avec l'Association des maires de France, que les associations d'élus étaient les plus à même d'épauler leurs édiles dans une bataille judiciaire, car elles sont capables de mettre à disposition leur expertise, ainsi que leurs ressources.

Actuellement, le droit en vigueur, au travers de l'article 2-19 du code de procédure pénale, ne permet qu'aux associations départementales affiliées à l'Association des maires de France d'intervenir pour les seuls élus municipaux. Je considère qu'il est impératif d'élargir ce dispositif aux associations nationales et à nos institutions, pour couvrir l'accompagnement de l'ensemble des élus, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux, nationaux ou européens. Le dispositif que je propose ne vise pas seulement les agressions physiques ; il permet également qu'une association nationale d'élus intervienne en cas de dégradation d'un bien d'un élu ou lorsque la victime est l'un de ses proches. Il prévoit aussi l'incrimination de l'exposition délibérée des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens. Il s'agit d'avancées majeures, attendues depuis des mois par les élus.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, mes chers collègues, la proposition de loi soumise à l'examen du Sénat s'inscrit dans la continuité de l'action menée par notre assemblée depuis déjà de nombreuses années.

Le texte qui nous est soumis répond également à une demande de l'AMF et rejoint les engagements pris par le Gouvernement en matière de protection des élus, notamment lors de la première version de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Il est important, je crois, de rappeler brièvement l'objet de l'article 2-19 du code de procédure pénale, que l'article 1 de la proposition de loi vise à modifier. Il s'agit, à l'origine, d'une initiative sénatoriale portée par nos anciens collègues Dinah Derycke et Michel Charasse en 1999. Ah, Charasse ! Son objet était de permettre aux associations départementales de maires de se porter partie civile en cas d'agression d'un élu. La plupart des associations départementales de maires interviennent, en effet, en appui financier, que ce soit pour payer les frais d'avocat ou les frais de justice, notamment la consignation au moment de la constitution de partie civile. Il était donc cohérent que ces associations puissent obtenir compensation en justice. Il me semble important de relever que la rédaction actuelle de l'article 2-19 vise les « instances introduites » par les élus. Seules, donc, sont concernées les affaires qui arrivent devant une juridiction. La constitution de partie civile dans le cadre de l'article 2-19 ne peut forcer à l'engagement de poursuites ou à l'instruction, et nous ne revenons pas sur ce point. L'Association des maires de France a, depuis vingt ans et tout particulièrement ces dernières années, développé son soutien aux élus victimes. Elle se substitue aux associations départementales lorsque cela est nécessaire. Elle a mis en place plusieurs dispositifs concrets d'assistance aux élus au cours des dernières années. L'inclusion de l'AMF paraît donc cohérente avec la possibilité, déjà ouverte pour les associations départementales de maires qui lui sont affiliées, de se porter partie civile. À notre connaissance, aucune autre association n'a mis en place de dispositif de ce type, à la fois adapté et discret. La volonté de Nathalie Delattre d'inclure, avec leur accord, l'ADF et Régions de France dans ce dispositif découle plus du souhait de permettre un soutien aux élus départementaux et régionaux et d'étendre ainsi à l'ensemble des élus locaux la faculté existant pour les maires. Nous n'avons donc pas souhaité, au stade de l'examen de ce texte par la commission, étendre au-delà de ces associations la possibilité de se porter partie civile, dans un souci d'efficacité et afin d'éviter toute concurrence entre associations et toute pression sur les élus.

à permettre aux collectivités territoriales et aux assemblées parlementaires de se porter partie civile en cas d'agression de l'un de leurs membres. Si la jurisprudence avait déjà admis une telle possibilité pour les assemblées, elle ne l'avait pas fait pour les collectivités, ce qui pouvait sembler incohérent. incohérent. Depuis la réunion de commission de la semaine dernière, nous avons poursuivi nos échanges avec le Gouvernement. L'esprit de compromis a finalement prévalu, et je tiens à saluer Mme la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et son cabinet, qui ont proposé une rédaction se rapprochant au mieux de l'objet premier de la proposition de loi et acceptée par la Chancellerie. La commission des lois a, en conséquence de cet accord, adopté un amendement qui vise à permettre à toutes les associations d'élus bénéficiant d'une ancienneté suffisante et répondant à des garanties statutaires et d'affiliation à une association nationale de se porter partie civile. Nous avons cependant tenu à reconnaître le rôle et l'implication de l'Association des maires de France dans la défense des élus municipaux. L'AMF, ADF et Régions de France restent donc expressément nommées, respectant ainsi l'esprit initial de la proposition de loi de Mme Delattre. Cet amendement tend également à réunir les articles 1 et 2 de la proposition de loi au sein d'un article unique, ce qui permet d'harmoniser les champs d'infraction et les personnes concernées, mais aussi de garantir la qualité juridique des termes employés. Nous sommes donc parvenus sur ce texte, me semble-t-il, à une solution susceptible de satisfaire une large majorité des acteurs. Cette proposition de loi apporte des réponses concrètes à certains dysfonctionnements dans l'accompagnement des élus et contribue à un exercice plus serein des mandats territoriaux et nationaux. Monsieur le garde des sceaux, madame la ministre, nous souhaitons qu'elle soit inscrite prochainement à l'ordre du jour des débats de l'Assemblée nationale

et les élus locaux sont, par leur engagement et le mandat qu'ils détiennent, les représentants de la démocratie nationale et locale. Ils occupent une place fondamentale dans le fonctionnement de nos institutions et, je tiens à le dire une nouvelle fois, toute atteinte à leur encontre, quelle qu'en soit la forme, constitue également une atteinte au pacte républicain. S'en prendre à un élu, c'est s'en prendre à la République. Ainsi que j'avais eu l'honneur de le souligner le 22 février 2022 lors de mon audition devant la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, le Gouvernement avait décidé, à la suite d'un intense travail avec M. Richard Ferrand, de permettre, dans un futur projet de loi, à la commune de se constituer partie civile, de même que l'Assemblée nationale ou le Sénat en cas d'infraction commise contre l'un Cela faisait suite à une violente agression qui avait touché le député Romain Grau à Perpignan, provoquant une vague d'indignation tout à fait légitime dans le pays. Au-delà de l'élu, nous avions également envisagé une telle possibilité en cas d'infraction commise contre sa famille, à laquelle on s'en prend parfois en raison de son lien avec l'élu. Je me réjouis donc de la proposition de loi que votre assemblée examine aujourd'hui. Dans la rédaction adoptée par votre commission des lois, elle rejoint un certain nombre de nos réflexions qu'il est indispensable de mettre en oeuvre. Malheureusement, les violences contre nos élus ne sont pas encore suffisamment endiguées. Depuis l'élection du Président de la République, nous recensons 509 affaires signalées d'atteintes aux élus ayant fait l'objet d'une transmission à la Direction des affaires criminelles et des grâces. Ces atteintes font désormais l'objet d'un suivi statistique très précis,

à obtenir des remontées fiables des parquets concernant les atteintes aux élus, dont j'ai fait l'une des priorités de ma politique pénale. Je suis donc en mesure de vous indiquer que, au total, 61 % des affaires concernent des faits d'atteinte aux personnes. Ce taux atteint même 80 % lorsque la victime est un maire. Néanmoins, le fatalisme en la matière n'est pas et ne et ne sera jamais de mise, et j'agis, avec ma collègue Caroline Cayeux, dont je veux ici saluer l'engagement, à nos niveaux respectifs, pour garantir une réponse pénale ferme, systématique et rapide. Depuis mon arrivée place Vendôme, j'ai cherché à tout mettre en oeuvre pour combattre, ou du moins mieux réprimer, les atteintes dont font l'objet nos élus. Car, disons les choses,

réside dans l'éducation des jeunes générations et l'apprentissage ou, plutôt, le réapprentissage collectif du respect élémentaire que nous devons à nos institutions. Toutefois, au-delà du civisme, il est de notre responsabilité à tous de ne pas banaliser ces actes insupportables et de les dénoncer, tous ensemble, pour ce qu'ils sont, à savoir des atteintes au pacte républicain. Si la justice ne peut réellement agir en amont, elle doit en revanche être très ferme, très efficace et très rapide en aval. Tel est mon rôle et celui de mon ministère, et nous l'avons, depuis deux ans et demi, pris à bras-le-corps. Par une circulaire du 7 septembre 2020, soit moins de deux mois après ma prise de fonctions, j'ai souhaité réaffirmer avec force l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre d'une politique pénale empreinte de volontarisme, de fermeté, de célérité et d'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales concernant les élus, afin qu'ils soient soutenus dans leur action quotidienne et qu'ils puissent la poursuivre sereinement. J'ai ainsi demandé aux parquets une réponse pénale rapide et systématique, en privilégiant les déferrements et, pour les faits les plus graves, la comparution immédiate. De même, un magistrat de chaque parquet a été désigné pour être l'interlocuteur privilégié des élus du ressort. Dans la circulaire du 15 décembre 2020 relative à la mise en oeuvre de la justice de proximité, j'ai demandé que soient réaffirmés le développement et l'approfondissement des relations partenariales avec les collectivités locales, le tissu associatif et les acteurs de terrain, afin de renforcer le dialogue institutionnel avec les collectivités locales et les maires. Voilà près d'un an, lors du Congrès des maires de France du 17 novembre 2021, j'annonçais à cet effet la création d'un groupe de travail visant à améliorer les relations entre les maires et l'institution judiciaire. Ce groupe de travail a rendu son rapport le 8 mars dernier, avec trente recommandations opérationnelles, parmi lesquelles j'en retiens plus particulièrement cinq sur le sujet qui nous préoccupe : améliorer la connaissance par les magistrats du ministère public de l'organisation des collectivités territoriales du ressort ; construire un partenariat avec les maires ; améliorer le dialogue entre les magistrats du ministère public et les maires ; accompagner le maire dans l'exercice de ses prérogatives en lien avec la justice ; enfin, développer la formation croisée des maires, des magistrats et de leurs collaborateurs. Ces préconisations entrent déjà, pour la plupart d'entre elles, dans les instructions de politique pénale générale que j'avais délivré aux parquets généraux dès mon arrivée Enfin, à l'occasion de la nouvelle circulaire de politique pénale générale du 20 septembre dernier, j'ai demandé avec force aux parquets de poursuivre le renforcement des échanges avec les élus, en premier lieu avec les maires et les présidents des conseils départementaux. La liste

ont fait l'objet d'une réponse pénale, et une poursuite a été engagée dans 92 % des cas. Quelque 114 condamnations ont été prononcées à ce jour, et une peine de prison l'a été dans 78 % des cas ; ce taux s'élève même à 81 % pour les cas d'atteinte aux personnes. Au-delà de la réponse pénale, il nous faut accompagner au mieux les élus victimes d'agression et les soutenir dans leur action judiciaire, en étant à leurs côtés tout au long de la procédure. Tel est le but de votre proposition de loi, madame la sénatrice Delattre, et je partage totalement cet objectif. Ce texte améliore les dispositions de l'article 2-19 du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction actuelle, n'autorise la constitution de partie civile qu'aux seules associations départementales affiliées à l'AMF, pour la défense des seuls élus municipaux et pour des infractions limitativement énumérées. Il élargit en particulier la faculté de se constituer partie civile à d'autres associations d'élus représentant divers échelons territoriaux l'Association des maires de France pour les élus municipaux, l'Assemblée des départements de France pour les élus départementaux et Régions de France pour les élus régionaux. loi reprend les dispositions précédemment mentionnées qui permettent aux assemblées d'élus elles-mêmes, ainsi qu'aux collectivités, de se constituer partie civile, y compris si la victime est un proche de l'élu. J'insiste à dessein sur ce point, car, si l'on dénombre, au 15 septembre 2022, quelque 509 affaires d'atteinte aux élus, ces affaires ont concerné 860 victimes au total. Il est donc urgent

exemple clair de la volonté de coconstruction législative qui doit guider notre action sur un sujet aussi crucial. Cet amendement a pour

des associations d'élus, qui sont désormais mieux définies et de manière plus équitable. Ainsi se trouve en particulier garantie la constitutionnalité du texte ; c'est bien le moins, me direz-vous

vous me l'accorderez, la désignation d'une seule association nationale, au détriment d'autres associations tout aussi respectables et légitimes.

tel regroupement permet de viser les mêmes infractions qui nous intéressent, à savoir tous les crimes et délits contre les personnes et contre les biens, certaines atteintes aux dépositaires de l'autorité publique et tous les délits de presse, dans une formulation claire et lisible pour tous les professionnels du droit. Il uniformise de surcroît la définition des proches des élus, en englobant à dessein les personnes vivant sous le même toit que l'élu, qui sont elles aussi, malheureusement, victimes d'agressions. Je le répète, les infractions commises contre les élus constituent à la fois des infractions contre leurs personnes et des atteintes à notre démocratie. Notre droit doit en tenir compte, en permettant que les élus soient officiellement soutenus au cours de la procédure pénale. En matière de lutte contre les atteintes aux élus,

Ces dernières années, nombre d'agressions, souvent médiatisées, ont servi d'alerte quant à l'exposition que consentent les titulaires de mandats électifs dans l'exercice de leurs fonctions. Il ne se passe pas une semaine sans que j'aie un contact avec un élu victime d'agression. Depuis le début de l'année, on dénombre une centaine de procédures, M. le garde des sceaux en a parlé : des procédures pour atteinte à l'encontre d'élus sont engagées chaque mois, concernant tous types d'atteinte, outrages, dégradations, menaces, violences.

cela avec pour unique but d'apporter aux élus la protection dont ils peuvent avoir besoin et qu'ils méritent. Il y va d'une exigence républicaine envers celles et ceux à qui nous devons tant, qui s'engagent pour le mandat qui leur est confié démocratiquement.

Le Gouvernement avait souhaité porter une disposition en ce sens dans la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur. Cela n'a pu se faire, mais notre résolution demeure inchangée. Nous sommes donc heureux de soutenir cette proposition de loi sénatoriale. texte vise à ce que, demain, les associations d'élus, telles l'AMF, l'ADF ou Régions de France, puissent se porter partie civile aux côtés des élus municipaux, intercommunaux, départementaux ou régionaux ou des membres les plus proches de leur famille.

équipées, puissent les accompagner en justice, afin qu'ils obtiennent la réparation qui leur est due lorsqu'ils ont été victimes d'une agression. Cette position, que l'AMF aussi défendait, se concrétise aujourd'hui au Sénat, dont on dit parfois qu'il est la maison des maires ou la chambre des collectivités. Les maires sont aux avant-postes, vigies de nos territoires, acteurs incontournables de notre vie quotidienne de citoyens et de responsables publics.

Le texte proposé va plus loin que les dispositions actuellement en vigueur, en ouvrant la possibilité aux associations nationales de se porter partie civile. Cette prérogative était jusqu'à présent réservée aux associations départementales des maires et s'agissant des seuls élus communaux. j'emploie le terme « possibilité », c'est que tout cela doit se faire dans le libre choix des acteurs : liberté des élus victimes d'agression de porter plainte et de demander le soutien de leur association d'affiliation, liberté des mêmes associations de soutenir les élus dans le respect de leurs capacités. L'élargissement du champ des associations concernées par la proposition de loi rejoint le souhait du Gouvernement ; je note qu'il fait consensus,

rencontrés par les élus. Dans le texte dont nous débattons, les élus peuvent être protégés contre toute diffusion d'informations visant à les mettre en danger.

Le champ des infractions s'étendrait aussi aux atteintes aux biens des élus. Cette mesure est nécessaire, comme l'illustre tristement le cas de l'incendie, en septembre dernier, du cabinet médical du maire de Saint-Pierre-des-Corps.

et les coûts qui résultent de leur obligation de protection fonctionnelle. La loi prévoit également que, dans les communes de moins de 3 500 habitants, le montant payé par la commune au titre de cette souscription fait l'objet d'une compensation

et de la justice était renforcée : les préfets signalent désormais systématiquement au parquet les faits dont les élus sont victimes et qui sont susceptibles de recevoir une qualification pénale. aux réponses pénales, elles vont dans le sens d'une plus grande sévérité et d'une plus grande fermeté, M. le garde des sceaux l'a rappelé. Vous le voyez, nous sommes au rendez-vous. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, ce débat au Sénat est une étape capitale : il doit être un début.